vous propose d'adopter une motion tendant à opposer la question préalable sur la proposition de loi relative au choix du nom issu de la filiation. Je le regrette très amèrement. Je le regrette d'abord pour toutes ces Françaises et tous ces Français qui placent leurs espoirs dans ce texte pour ces milliers de nos concitoyens qui vivent au quotidien la difficulté, voire la souffrance, de porter et même de supporter leur nom. Il ne tenait qu'à nous, Gouvernement Parlement, Assemblée nationale et Sénat, d'alléger ces difficultés, d'apaiser ces souffrances, par une réforme équilibrée et de bon sens. Je le regrette pour ces mères- de fait, c'est le plus souvent des mères qu'il s'agit -qui doivent justifier que leur enfant est bien le leur et présenter à tout bout de champ leur livret de famille. Je le regrette pour ceux qui ont hérité d'un nom qu'ils traînent comme un boulet. Je le regrette aussi pour le travail législatif, qui se trouve arrêté par ce qu'il faut bien appeler un front de conservatisme, malgré une recherche sincère de consensus avec M. Buffet, président de la commission Nous avons aussi pu compter sur le soutien d'un certain nombre de groupes de l'opposition, que je tiens à saluer. À gauche comme à droite, des efforts ont été faits pour trouver un compromis.

mais cela n'a pas suffi. Vos collègues députés ont fait le choix judicieux d'introduire un délai de réflexion pour le changement de nom dans le cadre de la procédure simplifiée, en prévoyant que le choix de nom soit confirmé devant l'officier d'état civil après un délai d'un mois au minimum. C'est là, assurément, une garantie que la volonté du demandeur est mûrement réfléchie et assumée. Malgré cela, non contente d'avoir détricoté purement et simplement ce texte en première lecture, la majorité sénatoriale refuse le débat.

dans le refus de voir la loi accompagner les évolutions de la société, je dis et je répète : vous faites fausse route ! Aux autres, qui attendent cette réforme, je dis qu'ils peuvent compter sur ma détermination et sur celle de l'Assemblée nationale pour faire aboutir le présent texte. N'en N'en déplaise à certains esprits chagrins, j'approuve totalement cette réforme, tout simplement par ce qu'elle répond à des attentes fortes de simplification. J'y insiste elle va faciliter la vie des mères et, au-delà, améliorer la vie de nombre de nos concitoyennes et de nos concitoyens qui supportent leur nom. Oui, mesdames, messieurs les sénateurs, cette réforme est juste.

si j'avais eu le moindre doute quant à l'utilité du bicamérisme dans notre République, ces deux années passées à vos côtés l'auraient dissipé

là, notamment dans la presse. Je serai tout à l'heure à l'Assemblée nationale pour permettre l'adoption définitive d'un texte qui fait oeuvre utile pour chacun de nos compatriotes.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, après l'échec de la commission mixte paritaire, nous sommes appelés à nous prononcer en nouvelle lecture sur la proposition de loi relative au choix du nom issu de la filiation, adoptée lundi par l'Assemblée nationale. Ce texte important, du point de vue tant des principes qu'il met en jeu que des conséquences qu'il peut avoir sur la vie de nombre de nos concitoyens et de leur famille, a été examiné en toute fin de session, avec une célérité qui ne me semble pas justifiée. Nous avons toutefois réussi à mener nos travaux avec sérieux et en faisant appel à l'expertise de nombreux professionnels : magistrats, avocats, personnels de mairie, pédopsychiatres, professeurs de droit, instituteurs, assistantes maternelles, C'est leur analyse qui a nourri la position de la commission, puis du Sénat, non des partis pris idéologiques, comme certains l'ont suggéré. Le Sénat n'a manifesté aucune hostilité à cette proposition de loi. il est conscient de la nécessité de simplifier les démarches de changement de nom pour répondre à certaines situations particulièrement douloureuses. Nous avons ainsi réussi à converger sur certains points, ce que nos collègues députés ont semblé oublier. nous avons accepté une souplesse accrue quant au nom d'usage, pour apporter une solution rapide aux personnes majeures qui souffrent dans leur vie quotidienne de devoir utiliser le nom d'un parent maltraitant ou délaissant. nous avons accepté une procédure de changement de nom simplifiée, sans justification d'un intérêt légitime, dès lors que le changement consiste à choisir un nom issu de sa filiation. accepté le principe suivant : donner aux adultes le même choix que celui des parents à la naissance de leur enfant, dans le cadre de l'article 311-21 du code civil, que ce soit pour leur nom d'usage ou pour leur nom de famille. Le Sénat a également adopté conformes l'article 2, qui donne compétence à la juridiction prononçant un retrait de l'autorité parentale pour se prononcer sur un changement de nom du mineur, et l'article 3, qui supprime l'intervention du tuteur pour un changement de prénom du majeur protégé.

divergence concerne la situation des mineurs, le second le rôle des communes. Toute notre réflexion a été construite autour de l'idée qu'un enfant ne fait pas la différence entre un nom d'usage et un nom de famille : le faire connaître dans sa vie de tous les jours sous un autre nom- c'est là le propre du nom d'usage, qui n'est pas une simple mention administrative -équivaut donc, en pratique, à lui faire changer de nom. De ce fait, l'article 1 de la proposition de loi présente à nos yeux un défaut de conception, puisqu'il repose sur l'idée qu'il serait

Nous avons été soucieux de ne pas perturber l'enfant dans la construction de son identité et dans sa vie sociale, dans un contexte conflictuel ou hors intervention du juge Nous n'avons pas souhaité autoriser une substitution de nom pour les mineurs à titre d'usage. Nous n'avons pas accepté non plus la solution proposée par nos collègues députés pour répondre à la demande de simplification exprimée par le collectif Porte mon nom. Le droit Porte mon nom. Le droit de décider seul, au cours de la minorité de son enfant, d'adjoindre à titre d'usage son nom de famille au nom de l'enfant, pourrait créer des situations instables : ainsi, l'enfant serait nommé différemment selon qu'il est chez son père ou chez sa mère et devrait revenir à son nom d'origine si le JAF considérait finalement qu'il n'est pas de son intérêt d'adjoindre l'autre nom. À l'article 1, le Sénat a donc préféré s'en tenir au droit existant pour les mineurs et maintenir la nécessité d'un accord des deux parents, s'ils exercent conjointement l'autorité parentale, ou d'une décision du JAF en cas de désaccord, ce qui est malheureusement fréquent. Les effets de la procédure de changement de nom simplifiée prévue à l'article 2 sur les enfants mineurs ne semblent pas avoir été suffisamment expertisés. Si l'on peut concevoir qu'un majeur puisse, une fois dans sa vie, choisir son nom par simple déclaration, sans aucune justification, il semble inopportun que ce changement de nom ait un effet automatique, par ricochet, sur les enfants de moins de 13 ans, sans aucun contrôle ni aucune information de l'autre parent. Notre second point de blocage concerne les communes. Nous n'avons pas souhaité que la simplification du fonctionnement du ministère de la justice se fasse au détriment des services de l'état civil des mairies. La procédure choisie dans le cadre de l'article 2 de la proposition de loi semble avoir été conçue de manière opportuniste pour pallier l'abandon d'un projet de numérisation et de dématérialisation de la procédure de changement de nom par décret, ainsi que les retards accumulés pendant la crise sanitaire.

Il s'agissait d'une procédure sur simple arrêté, et non plus sur décret du Premier ministre, que le ministère aurait engagée par téléprocédure sur la base d'un formulaire Cerfa. L'idée était de rendre cette démarche facile et accessible sur tout le territoire. Nous y avions apporté des garanties au moyen de l'institution d'une période de réflexion de trois mois et d'une recevabilité soumise à l'absence d'enfants mineurs pour éviter tout effet de ricochet. Cette solution n'a pas trouvé d'écho auprès des députés qui sont revenus à leur procédure initiale, sans autre changement que celui de prévoir un délai de réflexion d'un mois, ce qui semble insuffisant au regard de la portée de la démarche. Les députés ont donc peu ou prou repris l'intégralité de leur texte de première lecture. Ce n'est pas une surprise. Après le passage du texte au Sénat, ils ont aussitôt dénoncé un « détricotage », sans même relever les avancées votées par notre assemblée et que j'ai rappelées. Plutôt qu'un « détricotage », je parlerais d'un reprisage. Nous avons tenté, comme on le dit chez moi avec des mots un peu fleuris, de faire une robe de bal avec un sac à pommes de terre. Notre position a été présentée de manière caricaturale et le refus de toute évolution tendant à mieux prendre en compte l'intérêt de l'enfant et à ne pas transférer une tâche supplémentaire aux communes a entraîné une situation de blocage dont nous devons, malheureusement, prendre acte aujourd'hui. C'est pourquoi la commission des lois n'a pas adopté de texte et vous propose d'adopter une motion tendant à opposer au texte la question préalable. À cet instant, mon esprit vagabonde un peu, car je parle devant les statues de grands hommes d'État qui ont su faire des lois. Je pense à Antoine Blanc de Saint-Bonnet,

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, tout le monde n'a pas la chance de s'appeler Dupont et de naître en Normandie. Laissez-moi vous raconter ma petite histoire. Née à Istanbul, je suis arrivée en France en 1972, il y a cinquante ans déjà. Or les documents que j'ai pu produire au moment de ma naturalisation étaient ceux qu'Israël, où j'avais vécu sept ans, avait bien voulu me remettre. Les erreurs de transcription et de traduction aidant, je me suis ainsi appelée un temps Benbassat, avec un « t » final. Je me suis battue au fil des ans pour avoir un nom et un prénom qui soient vraiment les miens, mais le désordre n'a fait que s'aggraver. Je crus trouver la solution en arrachant un certificat de naissance à la Turquie et en le faisant transcrire en France. Hélas, en turc, je me nomme Ester, sans «

Mon nom et mon prénom continuèrent donc de varier selon les documents : passeport, carte d'identité, décrets de nomination, etc. Finalement, l'identité sous laquelle vous me connaissez ne fut longtemps qu'un nom de plume. En 2014, je décidai d'être moi-même une fois pour toutes. La bataille fut rude. En octobre 2015, je devenais enfin Esther avec un « h », comme l'héroïne

la seule graphie qui permette aux francophones de lire correctement mon nom, figurez-vous qu'il m'a fallu demander un changement de nom- que je finis, après cinquante ans, par obtenir en septembre 2016. Bref, je ne suis l'Esther Benbassa que vous connaissez que depuis cinq ans et demi, après presque un demi-siècle d'errance onomastique. Les motivations qui amènent qui amènent à entreprendre une démarche pour changer de nom sont, bien sûr, nombreuses, et touchent toujours à l'intime. Pensons à celles et ceux qui ont été victimes d'inceste, à celles et ceux qui ont été abandonnés par un parent, aux mères élevant seules leurs enfants, etc. Beaucoup trop de nos concitoyennes et concitoyens ne peuvent aller au bout

C'est regrettable. Je voterai contre cette motion.

texte : l'adjonction unilatérale, à titre d'usage, du nom du parent qui n'a pas transmis le sien, et une simplification réelle pour le citoyen de la procédure de modification du nom à l'état civil. C'est bien sur ces points que la majorité sénatoriale a opposé un refus de principe. Or cette réforme, attendue par les milliers de familles concernées, avait une utilité que personne, ici, n'a contestée. Il s'agissait d'une loi de liberté, puisqu'elle n'imposait rien à personne. Elle permettait tout simplement, d'abord, de donner aux mères la place qui leur revient dans le nom de leurs enfants, particulièrement dans le cadre des familles monoparentales. Elle soulageait ensuite la souffrance de nombreux citoyens souhaitant se détacher du nom d'un parent responsable de violences intrafamiliales, notamment après un féminicide ou un inceste. Elle représentait également un espoir pour nos concitoyennes et concitoyens qui portent le même nom qu'un terroriste, qu'un violeur en série, ou qu'un assassin tristement célèbre. Cette proposition de loi permettait, enfin, de faciliter les procédures administratives dont la durée et le coût représentent bien souvent des freins pour ceux qui souhaitent entreprendre les démarches nécessaires à un changement de nom. Ayant ces éléments à l'esprit, je dois avouer que je peine toujours à comprendre la majorité sénatoriale, qui semble avoir vu dans ce texte un énième coup porté au modèle familial traditionnel. Pourtant, il ne visait aucunement à invisibiliser les pères, mais bien à embrasser la diversité des situations familiales nouvelles, qu'elle concerne les familles recomposées, monoparentales, ou homoparentales. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, bien que perfectible, allait dans la bonne direction. Il nous appartenait de l'enrichir de nos propositions. Il aurait été de bon ton que, pour la dernière commission mixte paritaire de ce quinquennat, un esprit de concorde anime nos débats et règne Sur ce texte, je crains que la position majoritaire dans la Haute Assemblée ne réduise, hélas ! l'influence du Sénat. Aucun des apports dont nous aurions pu être à l'origine ne sera retenu, alors que notre rapporteur, Marie Mercier- que je veux saluer -et beaucoup d'entre nous avaient beaucoup travaillé pour améliorer cette proposition de loi. loi. Voyez-vous, mes chers collègues, ce qui me chagrine le plus, c'est que les Françaises et les Français qui attendent le vote de cette loi puissent penser, à tort ou à raison, que le Sénat a été insensible et sourd à leurs souffrances. Ils me l'ont écrit. Ils me l'ont dit. Cela me chagrine beaucoup- pour moi, et pour nous tous. Aujourd'hui, leurs regards et leurs espérances se tournent vers l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot dans le cadre de la navette parlementaire. Je ne doute pas que nos collègues du Palais Bourbon sauront adopter un texte répondant aux attentes exprimées. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, au moment de conclure mon intervention- la dernière de l'actuel quinquennat -, permettez-moi de vous saluer tous et toutes,

dont les dispositions devraient pouvoir entrer en vigueur en juillet prochain. Déposée par notre collègue député Patrick Vignal, elle a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale à une large majorité. à toute personne de modifier une fois dans sa vie son patronyme, de façon plus simple qu'il n'est possible de le faire aujourd'hui. En effet, si la procédure de changement de nom est d'ores et déjà possible dans certains cas- par exemple dans le cas d'un nom à consonance ridicule ou déconsidéré -, elle n'en reste pas moins difficile, coûteuse coûteuse et aléatoire. Il s'agit donc, d'une part, d'assouplir les modalités de changement de nom de famille. Tout majeur pourrait demander à prendre ou ajouter le nom de son autre parent. Cela pourrait se faire une simple démarche en mairie, sans justification. Je souligne que cette faculté demeurerait uniquement dans le cercle familial et ne permettrait en rien un choix totalement libre du nom. Il s'agit, d'autre part, de faciliter la vie des parents dont les enfants ne portent pas le nom. Ces situations fréquentes concernent en premier lieu les familles monoparentales et, par conséquent, très majoritairement les femmes. Ces dernières, à la suite d'un divorce par exemple, peuvent se retrouver contraintes de recourir systématiquement au livret de famille pour prouver leur lien avec leurs enfants lors de démarches banales : scolaires, administratives ou médicales. Pour sortir de ces situations, le texte de Patrick Vignal facilite pour les enfants le port, en plus du nom de famille donné à la naissance, du nom de l'autre parent au titre de nom d'usage. Nous sommes très favorables à cette évolution. L'objectif est de faciliter à la fois le quotidien des parents qui élèvent seuls leur enfant qui ne porte pas leur nom et celui des personnes majeures qui ne veulent plus porter le nom du parent qui leur a été transmis, pour des motifs affectifs- délaissement ou violences, par exemple. La procédure existante, par décret, est complexe et incertaine. Elle dure deux ans en moyenne et est soumise à de lourdes formalités de publicité. Au Sénat, le texte a été modifié de façon substantielle par l'adoption de plusieurs amendements. la suppression de la faculté de substituer le nom d'un parent à celui d'un autre à titre de nom d'usage de l'enfant, le maintien de la condition de double consentement pour procéder à une adjonction de nom, ainsi qu'une modification de la procédure simplifiée de changement de nom pour les personnes souhaitant porter le nom du parent Celle-ci ne se ferait plus directement devant l'officier d'état civil, mais devant la Chancellerie. La commission mixte paritaire n'est pas parvenue à une version de compromis. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli, en majeure partie, le texte initial. Toutefois, à l'article 2- qui est relatif à la procédure simplifiée susmentionnée -, les

Il est ainsi écrit que « le changement de nom n'est consigné qu'après confirmation par l'intéressé devant l'officier de l'état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande. » Nous sommes favorables à cette rédaction. Un certain nombre d'autres garanties sont prévues par ce texte. Elles ont été rappelées.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous regrettons que la commission mixte paritaire ne soit pas parvenue à s'entendre sur un texte commun. Nos deux chambres partageaient pourtant le constat essentiel suivant : la procédure actuelle de changement de nom est trop longue et bien trop complexe. L'Assemblée nationale, soutenue par le Gouvernement, proposait une simplification radicale. Par simple dépôt de formulaire, nos concitoyens auraient pu, une fois dans leur vie, changer de nom, adjoindre ou substituer à leur nom de famille celui du parent qui ne leur a pas transmis le sien. Le nom de famille est un héritage. Il nous est transmis sans que nous le choisissions. L'héritage est parfois bien lourd à porter. Certains noms sont des injures, d'autres finissent par le devenir. D'autres encore prêtent à rire, mais ne font même plus sourire ceux qui les portent. D'autres enfin renvoient à une histoire difficile et empêchent de tourner la page de violences ou d'abus. Celles et ceux qui souhaitent changer de nom de famille doivent saisir le ministère de la justice, puis justifier d'un intérêt légitime. Le changement nécessite la prise d'un décret et sa transcription. La commission des lois du Sénat convenait de la nécessité de simplifier la procédure. Elle proposait cependant de maintenir la procédure en vigueur, en la simplifiant. Les demandeurs qui souhaitaient changer de nom en utilisant le nom de leurs parents n'auraient pas eu à démontrer d'intérêt légitime.

était le maintien de sa solennité. La saisine du ministère de la justice en vue de la prise d'un décret et celle du Conseil d'État ne sont pas des démarches que l'on entreprend à la légère. Changer de nom n'est en effet pas un acte anodin. Certains de nos concitoyens craignaient un état civil « à la carte Nous comprenons ces préoccupations, fondées sur le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes. Cependant, rien ne nous permet de croire que nos concitoyens se saisiraient de cette possibilité à mauvais escient. La commission mixte paritaire n'a pas su s'accorder sur un dispositif commun. Les points de convergence étaient pourtant nombreux. Le Sénat souhaitait que les 3 000 à 4 000 demandes annuelles de changement de nom continuent d'être traitées par la Chancellerie. L'Assemblée nationale proposait quant à elle une procédure reposant sur les mairies. Nous comprenons parfaitement la logique consistant à décentraliser cette procédure et à la rapprocher de nos concitoyens. Il faut néanmoins rappeler que la durée moyenne d'une procédure de changement de nom est aujourd'hui de sept ans, alors que la procédure est gérée par le ministère de la justice. Un transfert de cette compétence vers les services municipaux entraînera nécessairement leur plus grande sollicitation. Une telle décentralisation doit être accompagnée des financements correspondants.

afin d'entendre, en application de l'article 18 de la Constitution, un message du Président de la République. En application du même article 18 de la Constitution, ce message ne donnera lieu à aucun débat. Par ailleurs, une déclaration suivie d'un débat, en application de l'article 50-1 de la Constitution, aura lieu la semaine prochaine, à la demande du Gouvernement. La conférence des présidents se réunira mardi 1 mars, à quatorze heures pour en fixer les modalités.

Toucher à l'institution du nom et à son évolution, c'est toucher à l'un des premiers marqueurs de l'identification d'une personne, mais aussi, indirectement, à son histoire personnelle, à ses origines et à sa descendance. Le nom évolue, change, disparaît parfois, fidèle en cela aux développements de nos vies humaines, traversées par des naissances, des mariages, des ruptures ou des décès. Modifier le droit des personnes ne peut ainsi se faire que prudemment, quelles que soient les douleurs vécues par tel ou tel.

Sur le fond, le Sénat a souhaité établir en première lecture un texte conciliant davantage stabilité du nom et volonté individuelle, afin notamment de mieux prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant qui a été le souci permanent de notre rapporteur, dont je salue le travail remarquable qu'elle a mené avec la sensibilité que nous lui connaissons. C'est dans un esprit constructif que notre assemblée avait suivi le Gouvernement à l'article 1 pour permettre aux majeurs la substitution d'un nom de Nous avions cependant refusé cette possibilité pour les mineurs, considérant que la substitution- qui va nettement plus loin que la simple adjonction -était un acte grave et que le droit existant s'avérait plus protecteur. Nous avions par ailleurs voté les dispositions de l'article 2 qui permettaient aux adultes, selon une procédure simplifiée, de choisir leur nom de famille parmi les noms issus de la filiation au premier degré, une fois dans leur vie. Nous avons été nombreux à reconnaître dans cette possibilité une mesure pertinente, à condition qu'elle ne soit pas banalisée sous prétexte de simplification administrative. Il nous faut, sur ce sujet, faire preuve de bon sens si la proposition de loi vise à faciliter le changement de nom, d'usage ou de famille, c'est bien parce que ses auteurs en ont reconnu l'importance symbolique et historique dans la vie de chacun. Comment, dès lors, envisager que l'évolution du nom puisse devenir un acte anodin, réduit aux plus simples formalités ? Nous en convenons tous, la procédure actuelle est dysfonctionnelle et lourde. Néanmoins, ce n'est pas parce que l'administration centrale fait face à une surcharge de travail qu'il convenait de se défausser sur l'échelon local. La proposition de loi envisageait une nouvelle procédure, déléguée aux communes. Nous nous y sommes opposés, tant pour maintenir la solennité d'une décision centralisée que pour éviter à nos communes de se voir confier une charge supplémentaire dont elles pourraient se passer. Nous avions proposé une procédure plus simple, conduisant à la prise d'un arrêté ministériel. Le Gouvernement s'y est opposé. Chers collègues, vous en conviendrez, les sujets de divergence avec le Gouvernement et la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale étaient nombreux et profonds. C'est à la fois la situation des enfants mineurs et la procédure décentralisée auprès des communes qui ont conduit à l'absence d'accord avec les députés lors de la réunion de la Nous constatons, pour le regretter, que le Gouvernement ne souhaite pas faire un pas en direction du Sénat. Les principales améliorations apportées par notre rapporteur n'ont pas été reprises par la majorité présidentielle. Monsieur le ministre, vous souhaitiez un texte consensuel et progressiste. Je constate que le consensus n'a été réalisé qu'entre vous et les députés de votre majorité, pour parvenir en fin de parcours législatif à un texte finalement bien peu enrichi.

Les dominations ne s'estompent pas d'elles-mêmes, il faut les contraindre à disparaître. Ce texte était une occasion de rendre la loi un peu moins sexiste, un peu plus juste, et de l'adapter aux évolutions de notre société. Un nom est bien plus qu'une convention sociale, c'est le symbole de notre individualité. Contraindre les femmes à y renoncer, c'est les invisibiliser. Les témoignages recueillis par le collectif Porte mon nom sont poignants. Que ce soit en raison d'une histoire douloureuse ou d'un nom difficile à porter, pour porter le même nom que ses frères et soeurs ou pour toute autre raison, changer de nom devrait être une formalité, une chose simple. Or que trouve la majorité sénatoriale à faire dans ces conditions ? Elle refuse l'ouverture de la substitution du nom d'usage dans le cadre de la filiation.

Elle refuse le changement de nom par formulaire dans les mairies, conservant la procédure incertaine, longue et opaque du décret ministériel. Elle refuse même de discuter une nouvelle fois tendant à opposer la question préalable, sous prétexte que l'Assemblée nationale ne reprend pas les propositions et les positions que je qualifierai de conservatrices défendues dans ce domaine par le Sénat. Dès la première lecture, nous avions fait état de nos inquiétudes face à ces positions et à leur justification. Décentraliser la procédure désorganisera les services des mairies, c'est une charge qu'il est déraisonnable de faire porter aux communes, dites-vous.

les divergences de points de vue entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur ce texte ont conduit à l'échec de la commission mixte paritaire. Certaines de ces divergences paraissant insolubles, les sénateurs de la majorité sénatoriale et Mme la rapporteure ont décidé d'adopter en commission une motion tendant à opposer au texte la question préalable, motion qui a été redéposée pour la présente séance par la commission des lois. Nous voterons contre cette motion, car nous partageons un certain nombre de points de vue défendus par nos collègues députés. De plus, nous étions favorables au texte initial et comptions sur la commission mixte paritaire pour qu'un accord favorable aux dispositifs initiaux soit trouvé. Si nous déplorons l'absence d'étude d'impact sur ce texte, nous pensons cependant que les 40 000 personnes qui ont signé la pétition à l'origine de ce texte ont de vraies revendications à faire valoir et que, pour accéder à la possibilité de changer de nom,

Je vous ferai grâce ici de mon histoire personnelle- ce n'est pas le lieu de la raconter. Un nom nous caractérise en tant que personne, mais également en tant que membre d'une famille, d'une généalogie, d'une histoire.

qu'on l'entend, qu'on le prononce ou encore qu'on nous demande de l'épeler. Le nom de famille peut être une ombre quotidienne dans le tableau de certaines vies. Mes chers collègues, il est déjà possible de changer de nom dans le cadre de la filiation. Toutefois, ce n'est pas certain, car cette possibilité s'accompagne d'une procédure de justification susceptible d'aboutir à un refus. Il est à nos yeux logique d'en faire un choix personnel indiscutable en simplifiant cette procédure. Pour ce qui est des mineurs, nous considérons que l'intérêt de l'enfant est parfaitement pris en compte dans la mesure où le texte vise simplement à donner au parent qui le souhaite, et qui rencontre des difficultés au quotidien pour prouver qu'il est bien le parent de son enfant, la possibilité d'ajouter son nom au nom d'usage de l'enfant. Si l'autre parent est absent ou s'il refuse de signer le formulaire de demande, aucun combat judiciaire ne devrait être nécessaire. L'argument selon lequel une délégation de la compétence à la mairie emporterait une charge supplémentaire ne tient pas non plus, à notre sens. Que la décision relève ou non du garde des sceaux, c'est à l'officier d'état civil qu'il revient de porter les changements sur les actes d'état civil dont disposent les mairies. Il paraît curieux, par ailleurs, de renvoyer le ministère de la justice à ses propres difficultés, que l'on sait grandes en matière d'outils numériques, et de lui demander de s'améliorer en conséquence. Enfin, sur le fond, on sait que les souffrances à l'origine d'une telle démarche s'inscrivent souvent dans un cadre d'inégalités entre les femmes et les hommes. Les femmes, mères, tributaires d'une histoire millénaire, donnent la vie à des enfants auxquels elles ne transmettraient pas leur nom et donc leur histoire familiale et une part d'elles-mêmes, au profit d'hommes, pères, qui, pour nombre d'entre eux, restent, parfois à leur corps défendant, ancrés dans des archétypes patriarcaux. Cette forme d'invisibilisation des femmes devrait désormais être révolue.

cette proposition de loi relative au choix du nom est attendue par certains de nos concitoyens, probablement plus que l'on ne l'imagine dans cet hémicycle. Quelle que soit la raison pour laquelle on en a besoin divorce qui se passe mal, souffrance liée au port du nom d'un personnage haï -, il est nécessaire d'améliorer la procédure, qui est aujourd'hui bien trop longue et dont le résultat n'est pas certain pour le demandeur. À l'Assemblée nationale comme au Sénat, nous partageons ce constat. Malheureusement, nos deux chambres sont en désaccord sur la méthode. Par exemple, s'agissant du nom d'usage, nous estimons que la substitution chez les mineurs soulève plus de problèmes qu'elle n'en résout, car substituer, c'est aussi un peu effacer ; or un enfant a besoin de ses deux parents pour se construire. Sur le nom de famille, ensuite, le texte prévoit un changement de la procédure. Nos collègues députés souhaitent expédier le changement de nom d'un coup de formulaire Cerfa ; il me semble que la position de la commission des lois du Sénat était plus mesurée, avec une amélioration de la procédure existante, en exemptant de toute justification d'un intérêt légitime une demande d'adjonction ou de substitution, pourvu que le nom soit issu de la filiation.

L'administration aurait largement eu le temps de s'améliorer, tant les problématiques liées à la procédure actuelle sont connues. Le Défenseur des droits avait tiré la sonnette d'alarme dès 2018, et l'informatisation du traitement des dossiers n'est toujours pas d'actualité. La simplification, La simplification, comme l'amélioration, aurait d'ailleurs pu être faite depuis longtemps déjà, la plupart des dispositions étant de nature réglementaire. Je ne peux que regretter une occasion manquée, surtout au regard du travail accompli par notre rapporteure, Marie Mercier, et du peu de divergences de fond qui nous séparaient d'un accord. Enfin, je rappelle que, pour qu'un dialogue, et donc une négociation, ait lieu, il faut que les deux parties soient ouvertes à la contradiction, ce qui n'a malheureusement pas été le cas sur ce sujet. En conséquence, au regard de ces divergences de fond comme de forme, le groupe Union Centriste votera la question préalable.

Je vous en épargne la liste. Toutefois, chacun comprend vite la portée de ce texte. Derrière un nom, se noue l'intimité des familles, souvent heureuse, mais, parfois, hélas ! dramatique. Derrière un nom, se retrouvent malheureusement certaines souffrances des enfants qui subissent les choix parfois brutaux de leurs parents ; ainsi de l'enfant élevé par un parent seul, mais qui se verrait imposer le nom de l'autre parent malgré son abandon, de l'enfant qui porterait le nom d'un parent maltraitant ou auteur de crimes contre lui,

Le droit actuel offre déjà des solutions, comme l'indique le code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom de famille. » Comme nom d'usage, toute personne peut utiliser un double nom, composé de son nom de naissance et du nom du parent qui ne le lui a pas transmis à la naissance. Aussi, pour chacune des deux situations, je vois mal quelle difficulté il y aurait à faciliter les changements dans les trois cas prévus : intervertir l'ordre de ses deux noms accolés choisis par ses parents substituer le nom de famille de l'un d'entre eux à son propre nom ; adjoindre à son nom, dans l'ordre que l'on choisit, le nom du parent qui ne l'a pas transmis. S'agissant du nom d'un parent, pourquoi faudrait-il justifier un tel changement ? Le travail des généalogistes dans les siècles à venir sera sans doute rendu plus difficile ; il n'en demeure pas moins que, avec ces dispositions, nous pouvons notamment soulager la souffrance d'enfants en leur donnant la possibilité de ne plus porter le nom de celui ou de celle qui fait de leur vie un cauchemar. Il est souvent question dans cet hémicycle de l'intérêt supérieur de l'enfant, quitte à y loger des considérations que les enfants ignorent eux-mêmes. Ce texte offre une authentique occasion de le défendre Vous comprendrez bien, mes chers collègues, que nous regrettions la position du Sénat. Certes, le choix du nom de famille n'a rien d'anodin et invite à la prudence. Aussi, j'entends le souhait d'éviter toute forme de précipitation lorsqu'il s'agit de jeunes mineurs, auxquels il faut garantir un cadre stable d'émancipation. l'avait toutefois souligné mon collègue Henri Cabanel, l'essentiel des dispositifs de cette proposition de loi ne prend rien à personne. Comme lui, je considère qu'il n'y a pas lieu d'infantiliser les citoyens. Le texte adopté par l'Assemblée nationale nous semblait équilibré et mieux à même de répondre aux problématiques soulevées. Au regard de tous ces éléments, mais aussi parce que, par principe, nous refusons que les débats s'arrêtent prématurément,

de vous avoir suffisamment exposé les raisons qui ont motivé le dépôt de cette motion. Il s'agit de prendre acte de la situation de blocage dans laquelle nous nous trouvons, malgré les avancées votées par le Sénat. Je tiens à remercier les collègues qui ont, pour

si la Chancellerie y consacrait les moyens nécessaires, elle pourrait garantir une procédure de changement de nom simplifiée, gratuite, sûre, rapide au lieu que celle-ci soit, comme aujourd'hui, difficile, coûteuse aléatoire et lente.

parfaitement improvisée a pour caractéristique principale de ne prendre en compte qu'une partie des personnes qu'il convient de protéger, et pas les autres. L'exemple vaut aujourd'hui pour les enfants : il me semble tout de même que

ou de conservatisme ; la modernité n'est pas plus une vertu que le fait de se rattacher à des principes fondamentaux. Monsieur le garde des sceaux, vous êtes allé trop vite et de manière trop simpliste dans cette affaire.

ensemble, aidé nos compatriotes qui le demandaient et que nous avions fait oeuvre utile. Ce n'était pas une grande polémique, monsieur le questeur. Vous savez quel point je vous respecte,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

d'abord assurer le peuple ukrainien de tout mon soutien et de toute ma solidarité.

; pas un sénateur ne mésestime ce que la France doit au monde combattant, à celui d'hier, à celui d'aujourd'hui et à celui de demain demain ; pas un parlementaire ne refuse d'échanger avec des associations du monde combattant ou de participer aux commémorations. Au-delà de nos appartenances partisanes, électorales prochaines et des divergences nécessaires au débat public, nous avons tous à coeur la reconnaissance et la transmission mémorielle. Nous tenons au soutien apporté par la Nation aux anciens combattants comme aux « nouveaux anciens combattants », ainsi qu'à la très grande diversité des ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre d'un engagement et d'un devoir de la Nation qui dépassent les générations. Nous sommes résolument attachés à maintenir le monde combattant comme maillon essentiel du lien armées-Nation. Nous affirmons notre volonté d'adapter les cadres du monde combattant à son évolution pour le pérenniser, pour le moderniser, pour qu'il fasse toujours écho chez les Français, pour qu'il soit toujours porteur des leçons et des valeurs auxquelles nous tenons : celles de la République. C'est la mission que je mène depuis près de cinq ans au sein du ministère des armées, c'est aussi le sens de cette proposition de loi. Celle-ci intervient à un moment clé de l'histoire du monde combattant,

; alors que, s'il rassemble encore plus de deux millions de femmes et d'hommes, le monde combattant se rétracte inéluctablement ; alors qu'il change de visage progressivement, avec la montée en puissance du nombre d'anciens des opérations extérieures, avec l'émergence de nouveaux profils de ressortissants, avec de nouvelles habitudes, de nouvelles pratiques, de nouvelles attentes. Dans cette perspective, j'ai veillé à ce que la maison des combattants qu'est l'ONACVG demeure l'opérateur principal du ministère des armées, qu'il reste un lien de proximité et un relais entre le monde combattant, la société civile et la puissance publique. À cet effet, je tiens à remercier sincèrement et chaleureusement, l'ensemble des équipes et des personnels de l'Office. J'ai eu plaisir à oeuvrer avec eux au cours des dernières années, à Paris comme dans tous les départements. Ces femmes et ces hommes accomplissent un travail remarquable au service de toutes les générations du feu, au service des pupilles de la Nation et des victimes du terrorisme, au service de nos blessés et de notre mémoire nationale. Changer le nom d'une institution plus que centenaire, ce n'est pas rien et ce n'est pas seulement symbolique. Cela a un sens éminent, la terminologie est toujours un message que nous délivrons aujourd'hui ensemble, résolument l'ONACVG vivra, le monde combattant a un avenir, les combattants d'aujourd'hui sont les héritiers des combattants d'hier et la Nation restera mobilisée pour accompagner et soutenir ceux qui servent sous le drapeau. La solidarité, la proximité et l'écoute resteront le coeur de l'activité et l'essence même de l'Office. Madame la rapporteure, je partage cette volonté, d'autant plus que le nouveau contrat d'objectifs

Cette longue vie, nous l'avons préparée au cours des derniers mois, avec le soutien inconditionnel des assemblées, avec l'application de la direction de l'Office, du conseil d'administration et de toutes les équipes nous avons oeuvré pour le maintien d'un service de qualité, pour l'accompagnement de la modernisation numérique ; nous avons engagé l'Office dans la dématérialisation, dans l'amélioration de ses instruments de relation avec les ressortissants, dans l'accessibilité numérique des prestations. Nous avons renforcé les services de l'ONACVG au sein des régiments, dans les espaces Atlas, en lien avec l'action sociale des armées. Nous avons sécurisé son action sociale propre dans la durée, en la professionnalisant encore davantage. Nous avons consolidé la solidarité et affermi la fraternité au bénéfice de tous les ressortissants, tout en maintenant le maillage départemental. Vous y teniez, j'y tenais : engagement tenu ! Nous le Nous le maintenons, car le lien humain et la proximité sont essentiels et les ressortissants en ont éminemment besoin. En matière de mémoire, nous avons confirmé

Avec l'ONACVG, nous avons constamment travaillé à la valorisation des nécropoles et au développement de l'innovation pédagogique sur les dix hauts lieux de la mémoire nationale. L'ONACVG continuera de creuser son sillon mémoriel, celui de la transmission de proximité avec une plus grande diversité de partenaires.

C'est à l'image de notre reconnaissance pour tous les combattants, de notre attachement au monde combattant et de notre volonté collective de faire vivre la mémoire. Exigence de la solidarité, passion pour la transmission : nous partageons avec fierté et sur tous nos territoires cette même ambition collective. C'est mon engagement et notre engagement commun pour la reconnaissance, l'attention et le respect que la Nation doit aux aux combattants qui l'ont servie.

présente proposition de loi, que j'ai déposée au début de l'année 2020- comme le temps passe vite ! -, a été adoptée par le Sénat le 9 mars 2021. L'Assemblée nationale l'a votée le 17 janvier dernier, complétée par deux amendements de coordination.

La volonté de modifier le nom de l'ONACVG s'explique par le fait que la population des ressortissants de l'Office ainsi que la nature de leurs besoins et de leurs attentes évoluent progressivement. Notre pays compte aujourd'hui près d'un million d'anciens combattants, essentiellement issus de la guerre d'Algérie. Cette troisième génération du feu, composée d'anciens combattants octogénaires, va, comme les deux précédentes, s'éteindre progressivement dans les années à venir. Lui succède depuis plusieurs années une quatrième génération du feu, composée des soldats engagés dans des opérations extérieures. S'ils justifient d'au moins quatre mois de présence sur un théâtre d'opérations, ces soldats peuvent bénéficier de la carte du combattant et relever ainsi des services de l'ONACVG. Ces hommes et, de plus en plus, ces femmes qui reviennent des théâtres d'opérations extérieurs peuvent donc être des anciens combattants et n'être âgés que d'une vingtaine d'années. Surtout, les besoins et les attentes de ces combattants sont bien différents de ceux de la troisième génération du feu. Étant plus jeunes, ils ont davantage besoin d'être accompagnés dans des projets de reconversion professionnelle ou de mobilité géographique. L'ONACVG s'emploie donc, depuis plusieurs années déjà, à diversifier ses missions pour amplifier ce type d'accompagnement. En effet, les missions d'accompagnement liées à la perte d'autonomie et aux invalides de guerre seront progressivement moins importantes à l'avenir pour l'ONACVG. Or, si l'Office adapte son activité aux besoins de ces « nouveaux » anciens combattants, ces soldats ne se considèrent pas tous comme des anciens combattants. Le nom même de l'ONACVG peut alors les dissuader de solliciter l'accompagnement proposé par l'Office, alors qu'ils en auraient besoin. Ils ne savent même pas forcément que cet accompagnement leur est accessible. Pour ces raisons, il est donc nécessaire que l'appellation de l'ONACVG soit mise en cohérence tant avec la diversification de ses missions qu'avec l'évolution de ses usagers, qui représentent le monde combattant dans sa diversité. Ainsi que je l'ai constaté lors de mes travaux sur cette proposition de loi et, plus largement, pour le monde combattant, il y a une attente forte de la part de cette quatrième génération du feu d'être davantage accompagnée et reconnue. Je crois que cette proposition de loi y contribuera. Elle constitue une étape dans les évolutions des politiques menées en faveur du monde combattant, lesquelles doivent s'adapter aux besoins de ceux qui se sont engagés pour notre pays. Ce changement de nom ne modifie ni les missions de l'ONACVG ni son organisation, laquelle se caractérise par un maillage territorial très utile pour l'accès de nos concitoyens aux services de l'Office. Il préserve également l'accompagnement déjà existant pour les anciens combattants et les actions de l'ONACVG pour la mémoire combattante. En somme, ce texte ne modifie donc que la désignation de l'ONACVG, pour que celle-ci soit mieux adaptée à la réalité du monde combattant et puisse accompagner les évolutions à l'oeuvre, qui sont liées aux nouvelles formes de conflit que connaît notre pays. Il propose ainsi de renommer l'Office, à compter du 1 janvier 2023, « Office national des combattants et des victimes de guerre ». L'examen en première lecture à l'Assemblée nationale a permis de compléter le texte par deux amendements de coordination, qui permettent de s'assurer que l'ensemble des appellations de l'Office qui figurent dans le droit positif seront remplacées par la nouvelle dénomination. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le Conseil d'État, l'organisation de l'ONACVG n'est pas parfaitement conforme aux règles de bonne gouvernance des établissements publics, car la loi prévoit aujourd'hui que l'Office est présidé par le ministre chargé des anciens combattants. Il serait en effet souhaitable de remédier à cette particularité frappée d'un risque d'inconstitutionnalité, afin d'éviter que l'autorité de tutelle ne soit également à la tête d'un établissement qui doit disposer d'une autonomie. des anciens combattants, que vous auriez souhaité compléter la proposition de loi pour résoudre cette difficulté. Toutefois, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec le texte tel qu'il a été proposé. Nous devons donc trouver prochainement un autre véhicule législatif pour sécuriser les règles de gouvernance de l'Office. Finalement, la commission des affaires sociales a approuvé la version du texte adoptée par l'Assemblée nationale. Elle vous propose donc, mes chers collègues, de voter cette proposition de loi sans modification, afin qu'elle puisse être définitivement adoptée. L'Office national des combattants et des victimes de guerre pourra ainsi développer ses missions d'accompagnement et de reconnaissance en faveur de l'ensemble du monde combattant. Enfin, en tant que présidente du groupe d'études Monde combattant et mémoire du Sénat,

Je vous remercie donc, madame la ministre, pour les échanges fructueux et respectueux que nous avons eus depuis 2018, et vous félicite pour l'ensemble des actions que vous avez menées en faveur du monde combattant au cours de cette période. Vous n'avez eu de cesse de consolider la reconnaissance de la Nation envers ceux qui l'ont servie avec passion et abnégation. Vous avez fait de la jeunesse un axe prioritaire de votre action, un point auquel vous savez que je suis attachée, et avez contribué à ancrer au sein de cette dernière les valeurs républicaines de solidarité, de fraternité, de citoyenneté- ce ne sont pas de vains mots ! -et de mémoire,

Engagée aujourd'hui en tant qu'auditrice au sein de l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), j'ai la chance de travailler aux côtés de jeunes colonels qui attendent impatiemment la promulgation de cette proposition de loi. Ce texte représente pour eux une réelle reconnaissance. La parole

je tiens en préambule à saluer le courage patriotique de tous ceux qui se sont battus ou qui vont encore se battre pour la sécurité de notre pays, ici ou à l'étranger. Je souhaite également remercier Jocelyne Guidez pour ce texte, que j'ai eu plaisir à cosigner avec ma collègue Gisèle Jourda. C'est effectivement pour la Haute Assemblée l'occasion de rappeler l'impérieuse nécessité, pour nous et pour les générations futures, d'honorer la mémoire des hommes et des femmes qui se sont sacrifiés pour la France, et pas seulement lors des commémorations officielles. Les actions de notre collègue Jean-Marc Todeschini, ancien secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, sont également à saluer, puisqu'il a contribué à sanctuariser les droits de tous les anciens combattants. C'est dans cette même logique de reconnaissance que le texte qui nous est proposé aujourd'hui a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale, après une légère modification rédactionnelle. Il s'agit donc d'harmoniser les dispositions législatives en remplaçant, à compter du 1 janvier 2023, l'appellation « Office national des anciens combattants et victimes de guerre » par celle d'« Office national des combattants et des victimes de guerre Cette modification sémantique symbolise politiquement non seulement notre attachement à cet opérateur public centenaire, que nous souhaitons voir préserver, mais aussi la prise en considération d'un monde combattant en mutation. les missions de proximité de l'ONACVG doivent être renforcées, car elles sont fondamentales. Grâce aux agents de l'Office et à toutes les associations bénévoles, les anciens combattants, mais également les pupilles de la Nation et les victimes du terrorisme, peuvent être accompagnés au quotidien, au plus près de leurs territoires. Cette dénomination marque aussi une volonté de modernisation, déjà développée par l'ONAC, et que nous devons continuer à encourager. En effet, les termes d'anciens combattants, en ne faisant référence qu'aux militaires ayant servi la France durant les Première et Seconde Guerres mondiales, occultent les militaires qui ont été engagés et qui le sont encore en opérations extérieures (OPEX), au Tchad, en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, dans l'opération Barkhane au Sahel et au Sahara, etc. Mon groupe est bien sûr favorable à cette stratégie d'adaptation, pour une plus grande reconnaissance des troisième et quatrième générations du feu, des soldats tués ou blessés lors de la guerre d'Algérie ou en opérations extérieures. Ce devoir de reconnaissance et de transmission de notre histoire commune est plus que jamais indispensable pour mieux vivre ensemble, et de façon pacifiée. Face à une population d'anciens combattants qui, inexorablement, se meurt, le monde combattant est amené à se féminiser, à se moderniser, à rajeunir, et se compose

nous en sommes conscients. Pour autant, mon groupe reste très attaché à ce que le service public délivré par l'ONACVG soit maintenu à un très haut niveau de qualité, ce que le maillage territorial, qui fait la force de l'Office, soit maintenu et renforcé. La présence de la centaine d'antennes et de services départementaux dans l'Hexagone et en outre-mer permet d'affirmer la continuité des grandes missions centrales de l'ONACVG, car nous demeurons catégoriquement opposés à toute tentative de régionalisation de l'Office. En effet, depuis septembre 2018, j'ai mis un point d'honneur à rencontrer toutes les associations d'anciens combattants et de victimes de guerre de la Guadeloupe, lors de réunions de travail, leurs difficultés. Je peux attester que la demande de proximité et de reconnaissance est bien réelle, tout particulièrement en outre-mer. Depuis les Depuis les dissidents antillais de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux Ultramarins ont toujours été présents sur les champs de bataille. Ce fut le cas de M. Octave

c'est dans un moment très particulier qu'intervient l'examen de ce texte, et je m'associe aux paroles de Mme la ministre sur l'Ukraine. Notre histoire contemporaine est le résultat du dévouement des fantassins, des tankistes de la ligne Maginot. Notre futur dépend du courage de ceux qui défendent, en ce moment même, les intérêts stratégiques de la France, mais aussi les valeurs et principes de la Nation. L'histoire du monde combattant, c'est tout simplement l'histoire de France. L'histoire du monde combattant a irréversiblement forgé une part de notre identité collective. Alors que nous débattons, de nombreux militaires sont engagés sur des théâtres d'opérations extérieurs. Je salue leur bravoure, leur engagement pour préserver la paix et les populations. J'aimerais également profiter de ce moment pour saluer la mémoire du brigadier Alexandre Martin, militaire du 54 régiment d'artillerie d'Hyères, mort il y a un mois à l'âge de 24 ans dans le cadre d'une attaque au mortier contre ce qui constituait la principale base de l'opération Barkhane, près de Gao. près de Gao. Bien évidemment, nous soutenons l'initiative de Jocelyne Guidez et de plusieurs de ses collègues, qui ont déposé cette proposition de loi. En visant à renommer l'« Office national des anciens combattants et victimes de guerre » en « Office national des combattants et des victimes de guerre crée ce trait d'union entre le passé, le présent et la transmission de la mémoire à notre jeunesse. Anciens combattants, militaires de l'armée française, victimes civiles d'actes de guerre ou de terrorisme, associations et fondations : ces acteurs constituent le monde combattant dans sa diversité, et ont toujours été écoutés par les parlementaires. Ici, au Sénat, nous nous accordons de manière transpartisane sur la nécessité d'une reconnaissance des droits à réparation et sur l'enjeu de la transmission de la mémoire. Je n'imagine pas une issue négative à ce texte qui correspond parfaitement à toutes les mesures mises en place sous ce quinquennat et votées par le Parlement. Je pense notamment au plan Ambition armées-jeunesse, présenté en mars 2021 et visant à renforcer les dispositifs existants en faveur de la citoyenneté, de l'attractivité et de l'égalité des chances. de finances pour 2022, qui a renforcé les droits des anciens combattants par une mesure d'ampleur touchant les pensions militaires d'invalidité et la retraite du combattant, et a également amélioré l'effort de solidarité en faveur des rapatriés, parmi lesquels, à titre principal, les supplétifs, leurs conjoints survivants et leurs enfants. Ainsi, 27 millions d'euros seront consacrés à ces personnes au titre des dispositifs actuels. Je me dois aussi de rappeler que le programme 169 de la loi de finances, « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation », a été renforcé par les actions concernant les liens armées-Nation, avec des crédits alloués à la Journée défense et citoyenneté, au service militaire volontaire ou encore aux politiques mémorielles. Je pense aussi à la hausse de 2 points de la retraite du combattant dans la loi de finances pour 2018, à l'attribution de la carte du combattant au profit des militaires déployés en Algérie entre le 3 juillet 1962 et le 1 juillet 1964, ou bien encore à l'extension de la reconnaissance des conjoints survivants des grands invalides de guerre. Madame la ministre, depuis votre arrivée au ministère des armées, vous avez répondu à nombre de demandes des associations jusqu'alors restées sans réponse. Ces mesures, ces dispositifs et cette proposition de loi ont une forte portée qui n'est pas que symbolique, et ils témoignent de notre attachement profond au système de reconnaissance, de réparation et d'accompagnement mis en oeuvre en faveur de ceux qui ont porté et portent encore nos armes.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nos forces armées sont engagées dans des opérations au dans la lutte contre le djihad, et contribuent à notre sécurité. Elles constituent la seule armée complète en Europe. J'aimerais saluer l'engagement extraordinaire des femmes et des hommes qui composent notre armée. Ils assurent la défense du territoire national, ainsi que la protection des intérêts de notre pays, au péril de leur vie. J'ai également une pensée pour les familles qui les soutiennent dans leurs engagements, mais aussi après le retour. La modification du nom de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre s'inscrit dans une volonté qui dépasse le changement de nomination. Cet office centenaire a pour but principal d'accompagner les anciens combattants ainsi que leurs familles. Tout au long de son histoire, ses missions se sont transformées au fur et à mesure des évolutions du monde combattant. Nous entrons dans une nouvelle phase de transformation pour l'Office et ses missions. Les objectifs restent cependant les mêmes et correspondent aux prérogatives de ce dernier : la reconnaissance et la réparation, la solidarité et la mémoire. Je profite du temps qui m'est accordé pour saluer l'action de l'Office et son implantation essentielle dans nos territoires. Chacun sait combien il est important d'aller au plus près de nos concitoyens. Ce texte, bien loin d'être symbolique, propose donc le changement de nom de l'Office dans toutes les dispositions législatives qui s'y rapportent. À ce titre, les modifications effectuées par les deux chambres du Parlement permettent de couvrir les différents codes et de revenir sur des erreurs d'appellation qui subsistaient dans certaines parties de ceux-ci. Je soutiens également l'évolution, depuis le dépôt du texte, intervenue en première lecture, ici au Sénat,

Je tiens à saluer le travail qui a été effectué tout au long de la navette parlementaire, et particulièrement ce qui a été fait au Sénat jusqu'à cette seconde lecture. La commission et notre rapporteure ont posé le cadre de débats constructifs. La paix n'est jamais acquise. Les tensions mondiales s'exacerbent et nous pouvons compter sur la volonté et l'action de nos forces armées. C'est inestimable et nous devons, nous aussi, leur apporter notre soutien. L'Office contribue à ce soutien. Nous devons lui donner des moyens suffisants pour remplir ses missions, et permettre un meilleur accompagnement de nos combattants, tout particulièrement pour ce qui est du retour à la vie civile. Ce point me paraît essentiel et il concourt aux évolutions multiples que nous vivons.

Nous examinons donc une seconde fois la proposition de loi relative au monde combattant. L'Assemblée nationale a jugé utile de modifier légèrement la rédaction du Sénat et en a profité pour corriger quelques incohérences entre les normes, ce qui ne change ni la nature ni l'objectif de ce texte que le groupe écologiste votera, comme en première lecture. Depuis maintenant plus d'un siècle, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre oeuvre auprès de nos combattantes, de nos combattants et de leurs familles pour leur apporter l'assistance et la reconnaissance qui leur sont dues. Pour assurer la pérennité et la mise en oeuvre de ses missions, l'ONACVG doit refléter une image fidèle de toutes celles et de tous ceux qui forment le monde combattant, afin qu'elles et ils puissent s'y reconnaître. Or, si aujourd'hui 30 000 personnes éligibles à la carte du combattant n'en ont pas fait la demande, si les associations du monde combattant peinent à fédérer la jeune génération, un constat s'impose : l'Office national des anciens combattants renvoie à un imaginaire collectif quelque peu dépassé. En effet, avec l'arrivée de la quatrième génération du feu, engagée dans des opérations extérieures depuis la décennie 1990, le monde combattant change progressivement de visage : il est plus jeune, plus féminisé, plus diversifié. Les membres de cette génération, moins nombreux que les anciens de la guerre d'Algérie, ont été engagés sur une plus grande variété d'opérations et ont un rapport exclusivement professionnel à leur service, très différent de celui des générations précédentes. Il est donc entièrement légitime que le nom de l'Office national chargé de leurs dossiers reflète cette évolution. C'est pourquoi le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires accueille favorablement la présente proposition de loi. Bien que ce changement de dénomination ne modifie pas les missions de l'Office, nous soutenons les initiatives visant à engager une réflexion sur le futur de la politique pour le monde combattant. L'entretien et la transmission de la mémoire des anciens combattants en sont des composantes essentielles, mais pas les seules. Si cette évolution ne s'accompagnait pas d'une attention supplémentaire aux besoins et demandes de ses nouveaux ressortissants, cette institution perdrait de sa pertinence. Cela se concrétisera notamment par des besoins accrus dans le domaine de l'accompagnement au retour à la vie civile et à la vie professionnelle ou par la reconnaissance des militaires engagés en opération intérieures. L'essentiel du travail reste donc à accomplir. Enfin, nous regrettons toujours l'abandon de la formulation originelle de la proposition de loi- Office national du monde combattant combattant -, qui permettait d'éviter le retour de la mention du genre des personnels de l'armée française dans ce nouveau nom. Si nous comprenons l'attachement au symbole qu'est le ONACVG ainsi conservé, nous regrettons que ce symbole contribue à perpétuer le peu de visibilité des femmes au sein de nos armées. une meilleure représentation des jeunes combattantes par l'ONACVG et par les associations du monde combattant s'imposent pourtant, particulièrement depuis le lancement du plan Mixité par le ministère des armées en mars 2019.

Plus de femmes, moins d'hommes : peut-être arriverons-nous un jour à l'équilibre ! Malgré cette réserve sémantique, et pour permettre une adoption conforme de ce texte avant la suspension, nous n'avons pas déposé d'amendement et nous voterons donc en faveur de cette proposition de loi. La

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi du groupe Union Centriste modifie l'intitulé de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, afin de tenir compte de l'évolution des conflits armés au XXI siècle. L'actualité ukrainienne illustre malheureusement la résurgence des menaces militaires dans le monde et sur notre continent. Notre groupe exprime, lui aussi, sa solidarité pleine et entière à l'égard du peuple ukrainien. En France, l'extinction progressive des générations entraîne une diminution du nombre d'anciens combattants qui représentent environ un million de personnes, pour l'essentiel des anciens combattants de la guerre d'Algérie. Le Sénat a adopté définitivement, le 9 février dernier, la loi portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie. Alors qu'auront lieu le 19 mars prochain les commémorations du soixantième anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, il est indispensable, dans un mouvement d'apaisement, de continuer le travail de mémoire des historiens et des chercheurs sur la colonisation et la guerre d'Algérie. Cette proposition de loi reprend une demande des associations tendant à moderniser l'image de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour attirer les jeunes militaires qui ne se reconnaissent pas dans la notion actuelle d'« ancien combattant En renommant l'« Office national des anciens combattants et victimes de guerre » en « Office national des combattants et des victimes de guerre », ce texte cherche à sortir l'Office de l'image négative de la notion d'ancien combattant. Cette modification est symbolique- beaucoup l'ont rappelé ici -, mais nécessaire, car le monde combattant n'englobe pas seulement les militaires qui ont servi la France lors des deux premiers conflits mondiaux, mais aussi de nombreux citoyens engagés sur des théâtres d'opérations extérieurs. Je pense notamment au Tchad, à la Côte d'Ivoire, au Liban, à l'Afghanistan, sans oublier nos forces mobilisées dans le cadre de l'opération Barkhane au Sahel et au Sahara. La reconnaissance des militaires dépasse le cadre sémantique ; elle prend aussi la forme d'une amélioration de la situation sociale et financière des personnes Alors que la réduction du nombre de bénéficiaires de la carte d'ancien combattant sert de justification, depuis des années, à la réduction des moyens de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour accomplir ses missions, il est impératif de réfléchir à l'amélioration de la prise en charge des combattants blessés, notamment les victimes Enfin, je voudrais rappeler le rôle indispensable des associations dans l'accompagnement social, financier et culturel des anciens combattants. Je pense en particulier à l'Association républicaine des anciens combattants créée en 1917 par Henri Barbusse et Paul Vaillant-Couturier, qui traverse actuellement des difficultés pour financer son journal. Le Gouvernement doit soutenir l'ARAC, comme toutes les associations, pour qu'elle poursuive son engagement centenaire en faveur de la lutte contre le fascisme, pour l'amitié et la paix entre les peuples, contre les inégalités et pour la défense de tous les droits sociaux. Les associations d'anciens combattants ne se contentent pas d'assurer

Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, chère Jocelyne Guidez, qu'il me soit permis, en ce jour où l'Ukraine a été réveillée par le bruit sourd de la guerre, de rappeler que la guerre est là, en Europe. Alors que j'ai une pensée pour nos combattants, nos héros et les victimes de guerre, je souhaite adresser le salut de la patrie au peuple ukrainien. Mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui en deuxième lecture la proposition de loi que notre rapporteure a déposée et qui vise à modifier l'intitulé de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, pour qu'il devienne l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Cette proposition a fait l'objet d'un consensus dès sa genèse : elle a été cosignée par de nombreux sénateurs au-delà de notre groupe centriste, après avoir été construite avec les associations du monde combattant et en lien avec le ministère. Je m'en réjouis. La modification de l'intitulé n'est pas qu'un symbole. L'auteure a proposé une modification qui tend, à la fois, à ne pas altérer la valeur de l'acronyme pour les anciens combattants et à permettre aux jeunes combattants de se reconnaître dans cet Office national. Je le rappelle, celui-ci délivre la carte du combattant à ceux qui ont servi au moins quatre mois, soit la durée d'une campagne d'OPEX, et leur propose un guichet d'accompagnement dès leur première mission. L'Office a bien pour objectif de s'occuper de tous ceux qui ont servi la France, qui ont choisi le métier des armes, ou encore les appelés qui ont servi sous les drapeaux. Nous parlons des anciens combattants tels que l'inconscient collectif les imagine je songe à ceux de la Grande Guerre, qui a fait 1,5 million de morts ou de disparus, à ceux de 39-45 ou encore à ceux des conflits plus récents d'Indochine et d'Afrique du Nord. Mais nous parlons aussi des anciens combattants des OPEX actuelles, ceux que l'on appelle la quatrième génération du feu. Je veux leur apporter tout mon soutien. Aujourd'hui, les anciens combattants d'Algérie, dont les plus jeunes approchent des 80 ans, sont près d'un million à être titulaires d'une carte du combattant selon les données des questionnaires budgétaires. Les guerres d'aujourd'hui ont changé de visage. Nos soldats se battent désormais sur les théâtres extérieurs, en OPEX. Nous débattions justement hier de l'implication de la France au Sahel. Comme l'exprime le Président de la République, ils sont « à la fois nos sentinelles et notre bouclier Les missions de l'ONACVG ne sont en rien modifiées par cette proposition de loi : reconnaissance et réparation, solidarité et mémoire. L'Office assure la reconnaissance de la Nation par l'octroi du titre de combattant et de la carte du combattant, qui compte actuellement un million de titulaires, un chiffre qui va malheureusement en décroissant. De plus, on estime à 30 000 le nombre de combattants qui n'ont pas demandé cette carte à laquelle ils ont pourtant droit. l'ONACVG assure l'accompagnement de ses ressortissants : vétérans des conflits et victimes civiles d'actes de guerre ou de terrorisme, mais également leurs descendants- pupilles de la Nation -et ascendants. Il assure, en complémentarité avec le ministère des armées, le retour à la vie civile et l'insertion professionnelle des combattants- des missions amenées à prendre une place croissante dans l'action de l'Office. Enfin, cette appellation combattante, active, permettra- je l'espère -de sensibiliser les jeunes soldats au devoir de mémoire envers les générations qui les ont précédés, mais aussi à la transmission de leur propre engagement auprès des jeunes générations et des associations et fondations pour entretenir et faire vivre ensemble cette mémoire dans les territoires. La mémoire des actions menées par nos militaires, leur engagement pour la France, parfois au péril de leur vie, péril de leur vie, constituent sans nul doute une composante importante de notre sentiment partagé d'appartenance à un grand État démocratique, en somme à l'idée que l'on se fait de la France. Cette proposition de loi sur la modification de l'intitulé de l'ONACVG est plus que symbolique, mais je crois à la force du symbole, car cette prise de position volontaire et engagée amorce une évolution nécessaire de la politique en faveur du monde combattant et, surtout, comme le souligne notre rapporteure, « impulse une évolution dans le regard que la société porte sur les vétérans des conflits ». Madame la ministre, nous n'ignorons pas que le Gouvernement souhaitait déposer lors de cette navette un amendement malheureusement irrecevable : il devait modifier les conditions de nomination du président du conseil d'administration du futur Office national des combattants et des victimes de guerre, qui est un établissement public à caractère administratif sous tutelle du ministre de la défense. Actuellement, la gouvernance de l'Office est assurée par « le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre Cette situation porte atteinte au principe d'autonomie de l'établissement public en plaçant l'autorité de tutelle à la tête de l'organe détenant le pouvoir de décision le plus général en son sein. Il faudra, à la faveur d'un autre texte, tirer les conséquences des remarques de la haute juridiction administrative pour que le président du conseil d'administration soit nommé par décret en conseil des ministres, à l'instar du directeur général. Soyez assurée de trouver trouver le soutien du groupe de l'Union centriste lorsqu'une telle modification sera présentée. Enfin, je salue le travail de coordination mené par nos collègues députés qui nous adressent un texte amélioré. Ainsi, notre groupe votera conforme cette proposition de loi qui, au-delà de l'intitulé, contribuera à renforcer la reconnaissance et le respect envers nos combattants, qui défendent, au prix de leur vie, nos valeurs et notre pays. La parole

ceux d'Algérie et d'Afrique du Nord, et ceux d'aujourd'hui, nos soldats en opérations extérieures : tout ce monde combattant, qui conjugue à la fois le passé et le présent, fait la fierté de notre pays. Je n'oublie pas le rôle particulier des forces supplétives en Algérie dont nous avons récemment discuté dans le cadre du projet portant reconnaissance de la Nation et réparation des préjudices subis par les harkis. Tous les sacrifices que ces catégories ont consentis pour la France justifient à la fois les hommages et les attentions. Depuis longtemps, l'État a mis en place une politique ambitieuse à l'égard du monde combattant déclinée par un volet mémoriel, d'une part, et un volet réparation, d'autre part. Régulièrement, au Sénat, nous tenons à l'enrichir, parce que, en tant qu'élus des territoires, nous recevons bien souvent le témoignage des combattants. Ce texte, qui vise à renommer l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, recueillera l'approbation du RDSE, car il répond à une attente, même si, fort logiquement, les combattants d'aujourd'hui seront les anciens de demain. Il traduit néanmoins une évolution, avec la disparition de ceux qui se sont engagés dans les grandes guerres ou les guerres d'indépendance. Ce qu'on appelle l'attrition naturelle ne doit en aucun cas conduire à l'oubli. Chaque année, le débat budgétaire nous invite à discuter des moyens de la politique de mémoire- M. Laménie le sait bien, puisqu'il en est le rapporteur spécial. Il est essentiel de les conserver afin de tenir éclairée la conscience de nos jeunes citoyens et de pousser certains d'entre eux à une forme d'engagement. Aujourd'hui, les anciens combattants ancrés dans notre imaginaire laissent la place aux soldats des opérations extérieures. Plus de Plus de 27 000 cartes ont été attribuées aux militaires ayant exercé leurs missions en Afghanistan. J'en profite pour saluer celles accomplies par les hommes et les femmes de l'opération Barkhane au Mali. Bien que la situation au Sahel soit encore très difficile, ils ont remporté des succès opérationnels qui méritent d'être soulignés, ne serait-ce que par respect pour les 53 morts pour la France et tous les blessés qu'il ne faut pas oublier. Au sein de ce nouveau monde, on le sait, il y a plus de femmes, plus d'actifs et moins d'invalides de guerre. Ce changement induit des besoins nouveaux, notamment en matière d'action sociale. Je ne doute pas que l'Office national des combattants et des victimes de guerre saura y répondre, tant que l'on préserve ses moyens et son maillage territorial. Madame la ministre, en tant que membre de la commission des finances, je suis heureux de voir que le contrat d'objectifs et de performance pour les années 2020 à 2025 de l'Office va dans ce sens. Mes chers collègues, de la première à la quatrième génération du feu, si le monde a changé, celui des combattants demeure, et la guerre n'est jamais loin, comme on le voit aujourd'hui en Ukraine, pays que nous soutenons bien Depuis toujours, ce monde représente un havre de fraternité, de mémoire et de solidarité, des valeurs qui nous sont chères et qui, au-delà d'un changement de nom, symbolisent la France, la patrie et la République.

Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, chère Jocelyne la proposition de loi que nous examinons cet après-midi va bien au-delà de la seule dénomination de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qu'il conviendra d'appeler, en 2023, « Office national des combattants et des victimes de guerre ». Elle nous permet d'avoir une réflexion plus globale sur le monde combattant. Avant de poursuivre mon propos, je tiens à saluer la mémoire de toutes ces femmes et de tous ces hommes, anciens combattants, qui ont sacrifié leur vie pour la France. Mes pensées vont également à tous nos soldats et à leurs familles, qu'ils soient en opérations extérieures ou sur le territoire national. Tous participent à notre sécurité, à la défense des valeurs de notre pays ainsi qu'à la paix en ces temps de graves troubles géopolitiques et de fortes tensions aux portes de l'Europe- et je tiens à m'associer à l'esprit de solidarité exprimé envers le peuple ukrainien - ; il importe de le mentionner. De la même façon, je tiens à rendre hommage à l'oeuvre des associations d'anciens combattants. Par leur action et leur mobilisation, ces associations ont construit, au fur et à mesure des décennies, un socle mémoriel pour notre pays et pour tous nos concitoyens, en particulier les jeunes. Honorer, préserver la mémoire, apaiser, unir, rappeler nos valeurs, transmettre les enseignements du passé, tels sont le rôle et les missions de ces associations. Qu'elles en soient sincèrement remerciées J'en viens maintenant à l'objet de la proposition de loi de notre collègue Jocelyne Guidez. Substituer les mots « anciens combattants » au profit de celui de « combattants » témoigne de l'évolution de l'état du monde et de notre société. Cela nous rappelle également combien la paix est précieuse et qu'elle n'est pas acquise. N'oublions jamais que l'Union européenne, c'est l'Europe de la paix. Comme cela a été précisé en commission des affaires sociales, ce texte doit permettre une meilleure reconnaissance des anciens combattants d'hier et de ceux d'aujourd'hui, et être l'occasion de rapprocher ces différentes générations qui ont en commun la fraternité d'armes et la défense du pays. Madame la ministre, un travail de rapprochement doit être mené entre les différentes institutions et les associations. Dans cette perspective, le rôle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est essentiel à différents niveaux. Cet organisme a évolué au fil des époques et des différentes générations du feu. En 1935, la fusion de l'Office national des mutilés et réformés, de l'Office national des pupilles de la Nation et de l'Office du combattant a donné naissance à l'Office national des mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de la Nation. C'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que cet organisme a pris son appellation actuelle. À ce jour, l'ONACVG intervient auprès des combattants et de tous ceux affectés par la guerre. Une politique de modernisation de l'ONACVG a été engagée il y a plusieurs années, elle se poursuit actuellement. Elle doit se faire également au bénéfice des veuves de guerre, des blessés de guerre et des pupilles de la Nation. Pour ce faire, l'ONACVG aura besoin d'un budget à la hauteur de ses missions et auquel nous continuerons d'être attentifs. Cette proposition de loi est une initiative bienvenue pour une meilleure reconnaissance de nos combattants d'hier et d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle le groupe Les Républicains votera en faveur de son adoption. La discussion générale

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture, à la demande du groupe Union Centriste, de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en première lecture, pour la mise en place d'une certification de cybersécurité des plateformes numériques

proposition de loi portant sur la mise en place d'une certification de cybersécurité des plateformes destinée au grand public. Cette proposition de loi, déposée par le sénateur Lafon, que je salue, le 15 juillet 2020, a fait l'objet d'une première lecture par les deux chambres,

À l'instar des évolutions numériques, dont nous devons nous réjouir, la cybercriminalité connaît malheureusement un essor sans précédent, les attaquants redoublant d'originalité pour détecter et exploiter nos vulnérabilités à des fins malveillantes. La menace cyber s'accroît, s'accentue et nous concerne tous, qu'il s'agisse des entreprises, des collectivités locales, des organismes publics comme des établissements de santé ou tout simplement des citoyens. Nous en avons eu de nombreux exemples ces derniers mois et années. La dangerosité des risques se mesure à la sophistication que les cyberattaques peuvent revêtir. Je peux ici citer l'hameçonnage, le, les logiciels espions, les virus, les faux supports techniques, etc. Les attaques cyber prennent des formes diverses et se démarquent par une capacité de renouvellement infinie. Nous avons par exemple vu exploser ces derniers mois le nombre des tentatives d'arnaque au compte formation. Cela dit, force est de constater que les choses évoluent et que ces risques sont mieux connus et mieux appréhendés. Depuis quelques années, un véritable chantier de pédagogie et d'information a été lancé, permettant à tous de prendre mieux conscience des méthodes utilisées par les cyberattaquants. Nous avons acquis avec le temps des réflexes d'hygiène numérique multiples, comme ne plus cliquer sur un lien envoyé par un expéditeur inconnu, ou encore faire des archives régulières de nos documents les plus importants.

Ces travaux visent à faire émerger des lignes fortes, solides et transnationales de nature à assurer au mieux notre souveraineté numérique. Comme pour le RGPD, l'Europe, en tout cas sa partie démocratique, doit se montrer à la hauteur des enjeux et définir ses propres standards. C'est pourquoi, face à ce panorama d'une menace cyber en pleine expansion, une adaptation de l'encadrement européen est apparue plus que nécessaire. Les institutions européennes sont donc en train de parachever la révision de la directive NIS, qui définit le niveau de sécurité des réseaux et des systèmes d'information au niveau européen. Nous soutenons l'approche ambitieuse de cette révision, puisque nous sommes convaincus que ces nouveaux standards de sécurité ne seront efficaces que s'ils s'appliquent à une échelle européenne. La deuxième réponse que nous devons apporter aux risques de sécurité- peut-être la plus importante, parce qu'elle est la plus « granulaire » et la plus systémique -est l'acculturation des utilisateurs, car l'information et la transparence sont des leviers décisifs du changement. Nous avons des exemples, désormais bien connus, de l'impact que la transparence et l'information peuvent avoir sur les comportements et sur les acteurs économiques. Le plus emblématique d'entre eux est peut-être celui de l'alimentation, auquel cette proposition de loi fait ouvertement référence.

La cybersécurité continue de pâtir d'une réputation de science froide, réservée à des utilisateurs avertis. Nous devons absolument lui retirer cette réputation et rendre accessible ce sujet crucial. C'est dans cette optique que vous proposez aujourd'hui l'établissement d'une symbolique visant à rendre clairement compréhensibles, pour les consommateurs, les enjeux découlant de la cybersécurité. Pour toutes ces raisons, je réitère évidemment le soutien du Gouvernement à la proposition de loi examinée aujourd'hui.

Les différentes lectures ont notamment permis de préciser les services numériques concernés et certaines des conditions dans lesquelles l'audit doit être réalisé et rendu public. Ces évolutions sont salutaires. Le législateur renvoie à l'exécutif le soin de préciser certains éléments plus subsidiaires. Nous nous y emploierons dans la continuité de l'état d'esprit constructif ayant présidé aux différentes lectures de cette proposition de loi- j'en remercie d'ailleurs les deux assemblées. La direction prise promeut une plus grande information du consommateur et une plus grande transparence de cette information. Sont ainsi posées les bases d'un cercle vertueux ayant fait ses preuves, ce qui sera très utile pour avancer vers une plus grande cybersécurisation des opérateurs. La parole

Cette initiative complète utilement les récents travaux du Sénat, en créant un dispositif qui se veut simple, lisible, et facilement compréhensible, pour informer les consommateurs du niveau de cybersécurité des principales solutions numériques qu'ils utilisent.

dans lequel il apparaît que 30 % des collectivités territoriales françaises ont été victimes en 2020 d'une attaque par rançongiciel, et que seulement 30 % d'entre elles ont par la suite mis en place un programme de prévention en cybersécurité. Si des efforts sont faits pour mieux informer les entreprises et les collectivités territoriales, nous constatons qu'aucune disposition législative n'oblige à informer les consommateurs sur les risques et le niveau de sécurisation des services numériques utilisés. Plusieurs législations nationales et européennes concernent la protection des données, mais les textes en vigueur sont finalement peu orientés vers l'information du consommateur. C'est donc ce manque que cette proposition de loi de notre collègue se propose de combler. Dans un quotidien de plus en plus virtuel, nous communiquons tous à l'aide de systèmes de messagerie instantanée, nous travaillons par l'intermédiaire de logiciels de visioconférence, nous nous informons en ligne en consultant les résultats de moteurs de recherche. Nous sollicitons aussi ces services pour nos usages privés : nous écoutons de la musique en ligne, nous nous divertissons sur les réseaux sociaux. Ces usages accrus du numérique ne vont malheureusement pas toujours de pair avec les pratiques et les précautions nécessaires. Les fuites de données, les piratages de comptes, les escroqueries en ligne, les attaques malveillantes et les failles dans la cybersécurité des entreprises, des hôpitaux, des collectivités ou des administrations sont de plus en plus fréquents. Si tous ces incidents nous sensibilisent chaque jour davantage aux enjeux liés à la protection de nos données, nos habitudes n'évoluent pas de pair.

ainsi que les logiciels de visioconférence, compte tenu de la généralisation de leur usage au cours de ces derniers mois. Après plusieurs modifications et de nombreuses hésitations du Gouvernement, la notion d'« opérateurs de plateformes en ligne » a finalement été retenue par l'Assemblée nationale. Le périmètre a été complété pour intégrer les systèmes de messagerie instantanée et de visioconférence, conformément aux souhaits de notre assemblée. Un deuxième enjeu concerne la nature et la dénomination du dispositif.

Un troisième point concerne le contenu de cet audit de cybersécurité, qui doit être défini par un arrêté ministériel. Sous l'impulsion du rapporteur de l'Assemblée nationale, et contre l'avis du Gouvernement, un amendement a été adopté afin de préciser que cet audit doit porter tant sur la sécurisation que sur la localisation des données. Une telle précision est importante, puisque la localisation permet notamment de déterminer le régime juridique applicable à la protection des données. Une localisation au sein de l'Union européenne implique la garantie de pouvoir bénéficier des protections permises par le droit de l'Union

Il nous semble donc essentiel que la Commission européenne prenne des décisions d'adéquation ou accepte des clauses contractuelles pour encadrer les transferts de données et attester que le niveau de protection est bien conforme ou équivalent à celui permis par le droit de l'Union, que l'hébergeur soit d'ailleurs européen

Ce point est crucial. Je rappelle que des données peuvent être stockées sur des serveurs et dans des centres de données localisées dans l'Union européenne, mais hébergées par des logiciels de américains. C'est toute la limite de la stratégie actuelle du label « de confiance » accordé à des entreprises qui utilisent également des licences de logiciels américains. Nous devons donc être vigilants et suivre avec attention l'élaboration de l'arrêté ministériel qui définira le contenu du futur audit de cybersécurité, afin de nous assurer que la localisation ne sera pas le seul gage

et compréhensible à l'aide d'un système d'information coloriel. Ces dispositions ont été maintenues sans modification à l'Assemblée nationale. Nous avions également supprimé l'article 2, qui modifiait les règles applicables à la commande publique

inédite et très technique. L'introduction de ce délai nous semble donc justifiée. Les mesures réglementaires d'application sont effectivement nombreuses. Le Gouvernement a indiqué que des consultations seront menées pour préparer cette élaboration.

Dans l'éventualité où des observations seraient formulées, le Gouvernement devant les transmettre au Parlement, les consultations liées à l'élaboration des mesures réglementaires d'application pourront donc permettre de prendre en compte les remarques de la Commission européenne et des autres États membres- nous y veillerons. Au-delà de ces points de vigilance et de ces précautions nécessaires, nous pensons à la bonne application de cette proposition de loi. Les modifications votées par l'Assemblée nationale nous semblent aller dans le bon sens et permettre d'atteindre les objectifs

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, ce début d'année 2022 constitue une nouvelle étape dans l'utilisation d'internet. d'internet. Depuis sa création, internet s'est révélé être un outil inouï tant pour l'innovation et la créativité que pour la saisie possibilités de progrès économiques. Indispensable, il participe à l'amélioration de notre qualité de vie, si bien que l'ONU veut garantir le droit à son

De plus, les risques cyber se multiplient nettement. L'Anssi a vu le nombre de cyberattaques traitées passer de 54 en 2019 à 192 en 2020.

n'a cessé de s'allonger. Face à cette nouvelle forme d'insécurité, il est important que les pouvoirs publics agissent davantage. Le Gouvernement s'est fixé des objectifs ambitieux afin de protéger la sécurité informatique des Français, et nous devons soutenir Afin de faire face à cette menace, un milliard d'euros seront mobilisés d'ici 2025, dont 720 millions d'euros de financements publics. Ces moyens permettront notamment de faire émerger trois « licornes » françaises en matière de cybersécurité, de diffuser une véritable culture de la cybersécurité dans les entreprises,

et des acteurs publics, afin de créer un environnement favorable à l'innovation technologique et au rayonnement de la filière cyber française. À terme, entre 1 600 et 1 700 personnes travailleront sur ce campus, dont 30 % représenteront les grandes entreprises et 25 % les services de l'État,

portera sur la sécurisation et la localisation des données. Enfin, cette proposition de loi est plus que jamais une réponse défensive face aux menaces cyber, car, au même titre que le Nutri-score, le Cyber-score permettra au grand public de savoir, en toute transparence, comment sont protégées les données personnelles.

collègues, une part de plus en plus importante de notre vie se déroule en ligne. Cette tendance s'est amorcée bien avant la pandémie, mais cette dernière n'a fait que la renforcer. De plus en plus de services sont dématérialisés : la banque, mais aussi la culture, ou même des consultations médicales.

Cette évolution présente donc de nombreux avantages, comme la rapidité, la facilité ou l'accessibilité, mais elle n'est cependant pas sans risques. Nous avons vu ces dernières années les attaques

sociétés commerciales se sont multipliées. Le dernier exemple remonte à quelques jours : des milliers d'informations personnelles des employés de Transavia, la filiale d'Air France, ont été piratées. Ces attaques nous rappellent à quel point nous avons besoin de protéger nos données. Le RGPD assure un haut niveau de protection des données personnelles des Européens à travers le monde.

Les sites internet les plus visités devront rendre publics les résultats d'un audit de sécurité, qui portera tant sur la sécurité de données confiées à la plateforme que sur la sécurité de la plateforme elle-même. Il s'agit donc d'évaluer le niveau technique de cybersécurité de ces sites. Ce dispositif nous semble particulièrement pertinent pour deux raisons. D'abord, l'approche technique nous semble indispensable aux côtés de la protection juridique. Ensuite, la publication des audits permet aux utilisateurs de bénéficier d'une meilleure information, afin qu'ils fassent des choix beaucoup plus éclairés, et qu'ils deviennent ainsi des acteurs de leur sécurité en ligne. Nous voulons dire à cet égard que l'Anssi ne remplit pas seulement un rôle d'expertise. Cette agence tient à développer les connaissances de nos concitoyens en matière de sécurité en ligne, car il s'agit d'une étape cruciale. Comme le remarquent de nombreux informaticiens, la faille de sécurité se situe souvent entre la chaise et le clavier. En devenant plus conscients des enjeux et des mécanismes du cyberespace, nous espérons que nos concitoyens deviendront plus exigeants. Ce texte constitue donc un réel progrès. Il nous rappelle également que nous devons bâtir la souveraineté de notre pays, y compris dans le domaine numérique. Nos données seront d'autant mieux protégées qu'elles seront hébergées sur notre sol, selon nos règles et sous la compétence de nos tribunaux. Le développement d'internet a affirmé la suprématie américaine dans ce domaine. Les dernières années nous ont démontré l'importance ultime de préserver notre indépendance et notre souveraineté numérique. Nous devons favoriser le développement de compétiteurs français. C'est à travers la concurrence que nous perfectionnerons les services et qu'une

traite un sujet capital, eu égard à l'importance toujours plus grande du numérique dans notre société et à la massification de son utilisation. Si le RGPD représente indéniablement une immense avancée en matière de protection des données,

Chacun d'entre nous a récemment entendu parler d'attaques informatiques contre des administrations ou des entreprises. Pas plus tard que le mois dernier, l'une des plus grandes villes de mon département a subi une attaque, et ses services informatiques ont été paralysés pendant plusieurs semaines. Outre les collectivités locales, le secteur de la santé et les entreprises sont aussi particulièrement visés par de tels types d'attaques. De nombreuses personnes sont conscientes de cette menace grandissante, et l'on s'attendrait à ce que tant les entités exposées à ce risque que les utilisateurs cherchent des solutions pour mieux protéger leurs données. Cependant, une réelle prise de conscience ne semble pas avoir lieu, malgré le fait que tout le monde s'accorde pour considérer que les données sont précieuses et doivent être protégées. Ainsi, si certaines entreprises, institutions et personnes sont bien évidemment vertueuses à ce sujet, nombre d'entre elles ont recours à des plateformes non sécurisées, qui ne garantissent ni une protection suffisante des données ni la confidentialité de ces dernières, ce qui les expose à de nombreux risques. Cette prise de risque a pour principale cause le manque d'informations quant au niveau de cybersécurité et de protection des données des plateformes.

Face à ce constat, il est indispensable que le législateur intervienne pour combler ces lacunes. Je remercie donc notre collègue Laurent Lafon de son initiative. Sa proposition de loi fixait deux objectifs améliorer l'information des utilisateurs de plateformes en matière de cybersécurité et sécuriser les données des acteurs publics, en faisant de la cybersécurité un critère supplémentaire lors des procédures d'appels d'offres pour les marchés publics. Le premier objectif se traduira par la mise en place d'un Cyber-score pour les plus grands acteurs du numérique, dans le but de mieux informer les consommateurs du niveau de sécurité des plateformes utilisées.

dans le cas contraire, l'objectif de cette loi ne pourra être atteint. Par ailleurs, puisque ce dispositif est entièrement à construire, nous devons être attentifs aux indicateurs retenus pour déterminer le Cyber-score d'une plateforme, car ces derniers peuvent être multiples et n'ont pas tous la même portée et la même signification quant au niveau de sécurité.

être proposées, qu'il s'agisse de la formation des entreprises à la cybersécurité, ou encore, comme la commission l'avait proposé, de la mise en place d'un crédit d'impôt à la numérisation des entreprises prenant en compte les dépenses visant à assurer leur sécurité informatique. Notre réflexion doit aller plus loin, car les enjeux liés à la cybersécurité et à la cybercriminalité ne feront que croître à mesure que notre société se numérisera. Mon groupe et moi-même voterons donc pour cette proposition de loi qui représente indéniablement une avancée. Mais j'invite encore une fois à pousser plus loin notre réflexion sur les questions de cybersécurité et de cybercriminalité,

Elle touche aux questions de la transparence et de l'information du consommateur internaute sur la sécurisation de ses données, ainsi qu'à la question de la souveraineté numérique tant en France qu'au niveau européen. En ce sens, nous remercions l'auteur de cette proposition de loi de mettre ce sujet si important Nous l'avions souligné lors de la première lecture : si l'évolution des technologies permet aujourd'hui une expansion du télétravail et peut simplifier les usages du quotidien, la cybersécurité est encore trop souvent sous-estimée. Sur ces enjeux, nous devons continuer de sensibiliser les citoyens, les entreprises ainsi que les collectivités territoriales et les pouvoirs publics, qui sont eux aussi souvent vulnérables aux cyberattaques. Nous devons rappeler que pratiquer le numérique, c'est aussi s'exposer à un certain nombre de risques. D'après l'Anssi, le nombre de cyberattaques a été multiplié par quatre en 2020. Face à ces actes, la question de la sécurité des systèmes est donc centrale. Si de nombreux textes régissent déjà la cybersécurité

Nous soutenons ainsi la principale mesure de ce texte, la mise en place d'un Cyber-score, c'est-à-dire d'un diagnostic de cybersécurité lisible, clair et compréhensible par toutes et tous. Je m'interroge néanmoins quelque peu sur la portée du texte. Si, à la suite de la navette parlementaire, le champ d'application du dispositif est étendu à tous les services numériques, notamment aux logiciels de visioconférence et de messagerie instantanée, également limité aux services numériques les plus utilisés, selon des seuils définis par décret. Renvoyer ainsi au pouvoir réglementaire l'établissement de la liste des plateformes concernées par cette obligation de communiquer les informations relatives à la sécurité des données hébergées risque de limiter la portée du dispositif. Pour garantir une réelle efficacité de la mesure, il faudra que le décret ajuste au mieux les mailles du filet, afin de ne pas exclure de nombreuses entreprises du champ d'application Si la commission et l'Assemblée nationale ont justifié cet aménagement pour éviter d'imposer « de trop fortes contraintes à de petites structures », nous pensons au contraire que les petites entreprises du numérique ont tout à gagner à faire valoir la fiabilité de leurs plateformes et à faire respecter une gestion responsable Concernant les apports adoptés par l'Assemblée nationale, nous saluons certaines dispositions. Le périmètre de l'article 1 a été élargi afin d'inclure les systèmes de messagerie instantanée, en plus des logiciels de visioconférence. L'audit devra être réalisé par des prestataires agréés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et devra porter sur la sécurisation et la localisation des données.

C'est pourquoi, comme l'a souligné Mme la rapporteure, le Parlement devra être vigilant dans les mois à venir sur l'élaboration de ces mesures. En définitive, malgré ces quelques points non négligeables, avec cette proposition de loi, le Parlement pose une première pierre et apporte une contribution utile au renforcement de la protection des données de nos concitoyens. Nous voterons donc de nouveau en faveur de ce texte. La parole

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, comme nous l'avions dit en première lecture, cette proposition de loi est bienvenue, car aujourd'hui aucune disposition ne garantit l'information du consommateur et de la consommatrice quant à la sécurité informatique de la solution numérique qu'il ou elle utilise. En ce sens, ce texte représente un pas supplémentaire vers davantage de transparence et de droits pour les internautes. À l'ère où l'informatique, omniprésente, pénètre tout notre quotidien, la question de la sécurité des systèmes reste centrale. d'un enjeu essentiel tant pour l'économie que pour la démocratie. En effet, l'outil proposé permettra un accès plus facile aux problématiques et enjeux de la cybersécurité,

Aussi, la mise en place d'un Cyber-score calqué sur le modèle du Nutri-score, qui concernera, outre les plateformes en ligne, les logiciels de visioconférence et les systèmes de messagerie instantanée, est une bonne chose. Autre point positif : le système d'autoévaluation des entreprises concernées. Le principe d'une contrainte plus lourde a été adopté par l'Assemblée nationale et maintenu par la commission des affaires économiques du Sénat : il s'agit de l'audit de sécurité qui devra être réalisé par des prestataires agréés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et qui portera tant sur la sécurisation que sur la localisation des données. Les résultats de cet audit devront être présentés au consommateur, pour les informations relatives tant à la sécurisation qu'à la localisation des données hébergées. Nous l'avions mentionné à plusieurs reprises,

occuper aujourd'hui. Les nouvelles technologies se sont invitées dans les foyers des particuliers, toutes générations confondues. Cela s'est bien évidemment accéléré avec la pandémie de covid-19 : il s'agissait en effet de trouver de nouveaux moyens de communication pour entretenir le lien social, s'informer, se divertir. Selon une étude récente, aujourd'hui, près de 50 % de la population mondiale utilise les réseaux sociaux. Pourtant, malgré une médiatisation accrue des sujets liés à la cybersécurité ou aux- ces fameux logiciels malveillants ciblant les particuliers et les entreprises

de la sécurité informatique et de la cybersécurité. Les entreprises ont bien perçu les énormes risques économiques auxquelles elles peuvent être confrontées en étant piratées, espionnées ou sabotées.

La prise de conscience des entreprises et des organisations publiques est essentielle, car les cyberattaques les visant présentent un risque réel pour le grand public, en mettant en péril les données personnelles de milliers de clients ou d'utilisateurs. une pédagogie sur les risques numériques, rappeler que la cybersécurité est désormais l'affaire de tous, tout cela relève, en quelque sorte, d'un enjeu citoyen qui doit être au coeur de nos préoccupations. En ce qui concerne les usagers, selon une enquête récente, 96 % des Français interrogés sur le sujet se disent conscients que l'usage des outils numériques comporte des risques. Pourtant, ils reconnaissent ne pas avoir intégré ces risques

à des vidéoconférences ou encore à télécharger des contenus risqués. Chacun confie, dans son quotidien, par un simple clic, plus ou moins volontairement, de nombreuses données personnelles qui sont ensuite stockées, utilisées, traitées et même vendues par les plateformes numériques qui les gèrent. La sécurité de ces données est essentielle. Les usagers ont besoin de solutions simples et accessibles pour être informés des risques encourus et pour se protéger. Or, à ce jour, aucune disposition ne garantit l'information du consommateur quant à la sécurité informatique de la solution numérique qu'il

de bien en définir les critères et surtout de les adapter aux évolutions des plateformes et des usages des particuliers. L'enjeu est pour nous de construire un monde numérique plus sûr.

enjeu de longue date et pourtant sous-estimé, est encore plus cruciale depuis la mise en oeuvre des mesures de lutte contre la pandémie de covid-19 et le recours massif aux outils numériques dans le cadre du télétravail, des besoins courants ou encore des loisirs, sans parler de la montée générale des tensions nationales et internationales. On ne peut que regretter un certain retard français en matière de culture de cybersécurité, comme l'a rappelé récemment le directeur de l'Anssi devant la commission des affaires économiques. La nécessité d'informer le public et de lui donner des outils concrets est donc réelle. Face aux risques de piratage ou de cyberattaque, nous sommes tous vulnérables : individus, consommateurs, mais aussi entreprises, institutions ou collectivités. Dans ce contexte,

Le contenu de ce texte a quelque peu évolué depuis sa version initiale : inclusion des téléconférences dans le champ d'application de la certification, compétence explicite de l'Anssi pour qualifier les prestataires remplacement du diagnostic de cybersécurité par un « audit », selon la terminologie actuelle. Plus cruciale sans doute est l'inclusion de la localisation des données hébergées par les plateformes, qui est, nous le savons, un fort enjeu de sécurité et de souveraineté numériques.

comme son équivalent alimentaire, peut receler des situations hétérogènes. Un enjeu majeur du texte- le périmètre des plateformes concernées par la certification -est toutefois définira un seuil de déclenchement. Souhaitons que ce seuil permette de viser les plateformes les plus répandues sans pour autant pénaliser les PME et les start-up. Enfin, l'article 2 qui concernait initialement les appels d'offres dans le cadre de marchés publics a finalement été supprimé. Ainsi, cette proposition de loi, pour utile qu'elle soit, n'est qu'un début, puisqu'elle nécessitera des mesures réglementaires, d'où une entrée en vigueur finalement repoussée au second semestre de 2023. Elle devra aussi trouver sa place dans le cadre européen défini par le règlement général européen sur la protection des données personnelles. Notre groupe votera pour son adoption, comme il l'avait fait en première lecture, tout en gardant à l'esprit les défis à venir.

nous examinons en deuxième lecture la proposition de loi visant à mettre en place une certification de la cybersécurité des plateformes numériques. Au cours des dernières années, plusieurs affaires ont éclaboussé le monde de l'industrie numérique, avec d'importants faits de fuites et d'exploitation de données personnelles. particuliers ou à des entreprises, les données stockées dans le cyberespace ont été la proie d'attaques qui se sont multipliées à un rythme quasi exponentiel au cours des dernières années, tandis que les solutions numériques proposées sont de plus en plus complexes, raison d'algorithmes toujours plus puissants et toujours plus opaques. Les acteurs de ce marché développent de nouveaux usages, fondés sur l'analyse de nos données personnelles,

La crise sanitaire que nous subissons et dont nous peinons à sortir a amplifié ce phénomène. En raison des confinements répétés que nous avons traversés, la dématérialisation de notre société a été accentuée, accélérée, alors que, dans le même temps, la relation de confiance entre les citoyens internautes et les géants de cette industrie s'est dégradée, sans que cela remette en cause l'hégémonie

Malheureusement, les événements tragiques qui se déroulent à l'Est, auxquels de nombreux collègues ont déjà fait référence- je m'associe d'ailleurs à ces derniers pour condamner ces attaques et exprimer mon soutien au peuple ukrainien

CSNP avait recommandé aux pouvoirs publics de développer une politique massive d'information et de sensibilisation de la population aux risques encourus dans l'espace numérique, à titre tant privé que professionnel, et de prendre les mesures et dispositions permettant de s'en prémunir. Ces alertes rejoignent celles qui figuraient dans le rapport de la commission d'enquête sur la souveraineté numérique, présidée par notre collègue du groupe socialiste Franck Montaugé : « Dans un univers numérique marqué par une forte asymétrie entre, d'un côté, ceux qui contrôlent données et algorithmes et, de l'autre, ceux qui utilisent les plateformes, imposer le respect de ces droits et les rendre effectifs pour les particuliers reste encore concrètement à accomplir. » Je me réjouis donc de voir le législateur se saisir de ce sujet. Nous devons être à la hauteur des enjeux que recouvre la question de la cybersécurité. La garantie de la protection de la vie privée de nos concitoyens est une des garanties clés de notre démocratie. La mise en place d'un Cyber-score va dans le bon sens, sous réserve que l'État s'en saisisse pour sensibiliser massivement la population à ce sujet. Veillons à ce que le développement et l'essor du numérique soient toujours synonymes de l'émancipation des femmes et des hommes et non de leur aliénation.

en stockant du fourrage lors des bonnes années pour faire face aux mauvaises et en inventant l'irrigation pour lutter contre la sécheresse ou le drainage pour lutter contre l'excès d'eau,

Ce sujet m'imposait de ne pas faire de politique politicienne. Sans esprit partisan ni arrière-pensée, j'ai travaillé à la

par la possibilité de lutter contre les injustices flagrantes du système indiciel, par l'institution d'un droit de recours collectif et par

au sujet si important de l'assurance récolte. C'est vrai, mesdames, messieurs les sénateurs, vous étiez d'accord sur le fond avec cette réforme. D'ailleurs, vous aviez pleinement conscience de la nécessité d'avancer sur cette question, puisque le Sénat participait à cette réflexion depuis

encore sur un quatrième principe, celui de la régulation, avec la constitution d'un pool mutualisant les risques, l'élaboration d'une tarification technique commune et une plus grande transparence dans la constitution des prix.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je crois pouvoir dire, en toute humilité, que vous allez aujourd'hui voter une réforme historique, fruit d'un travail parlementaire toujours

Le changement climatique met à lourde épreuve notre agriculture ; il fragilise son économie et notre souveraineté alimentaire. Le projet de loi portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture était, comme je l'ai déjà dit, extrêmement attendu par les acteurs du monde agricole. Sa nécessité n'est pas à prouver. Je tiens tout d'abord à féliciter la commission et notre rapporteur de leur travail. Je veux aussi vous remercier, monsieur le ministre, pour votre constance et votre implication sur ce dossier ô combien important pour nos agriculteurs et pour notre souveraineté alimentaire. Ce projet de loi a été conçu au plus près des acteurs du milieu afin de répondre à leurs besoins. Il refonde toute la politique d'accompagnement assurantiel et de gestion des risques climatiques en agriculture.

Il nous fallait renouveler les outils dont nous disposions, de moins en moins adaptés et souvent inopérants au regard de la fréquence et de l'intensité des aléas climatiques et de l'évolution de notre agriculture.

En effet, les offres assurantielles devraient être plus attractives et plus incitatives. Le Sénat s'est attaché à lever les freins à la souscription grâce à la minoration de la prime, la préservation d'un droit de contestation pour les évaluations des pertes et à la révision des surfaces minimales à couvrir dans les contrats. Le soutien européen

compris dans un subventionnement fixé à 70 %. Enfin, l'État interviendra dès 30 % de pertes dans les filières les moins assurées. Ce texte prévoit un réel accompagnement de l'État grâce au soutien financier important de la solidarité nationale qui passera de 300 millions à 600 millions d'euros par an en moyenne. Enfin, la dernière avancée majeure que je tiens à souligner réside dans la mutualisation des risques et la constitution de ce pool d'assureurs afin de construire et de garantir un produit homogène et universel.

au coût de cette réforme. Les arbitrages sur le financement ne font pas l'objet de dispositions budgétaires précises. Tout est donc renvoyé au projet de loi de finances pour 2023 et à des dispositions réglementaires qui seront prises ultérieurement. Néanmoins, il est indéniable que la gestion des risques climatiques ne peut uniquement reposer sur l'attractivité de l'offre assurantielle. D'autres leviers et éléments essentiels doivent être mobilisés mobilisés : technicité de l'agriculture, recherche et innovation, évolution des pratiques, constitution de stocks, meilleure gestion de l'eau et épargne de précaution. Ce texte, qui porte aujourd'hui la marque du Sénat, bâtit un cadre législatif équilibré et garantit aux agriculteurs une lisibilité sur l'outil de gestion des risques. Bien évidemment, le groupe Les Indépendants votera avec enthousiasme en

de souffle. Les deux systèmes qui cohabitent actuellement- indemnisation publique en cas de calamité agricole et aide à la souscription d'un contrat d'assurance -laissent sans réponse des pans entiers de notre agriculture.

ailleurs, la fréquence et l'intensité des aléas climatiques auxquels sont confrontés les agriculteurs menacent l'équilibre financier du dispositif actuel. Nous avons tous en tête le fort épisode de gel du printemps 2021, pour lequel l'État a dû exceptionnellement débloquer 1 milliard d'euros et rendre éligibles aux indemnisations les zones viticoles touchées. Nous nous réjouissons surtout de voir que les apports du Sénat ont été maintenus dans le texte final. Il s'agira, demain, d'une loi d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture. Je veux saluer le travail de la présidente de la commission des affaires économiques, Sophie Primas, et celui de notre rapporteur, Laurent Duplomb, qui sont parvenus à donner corps à l'architecture initiale, parfois imprécise, que proposait le Gouvernement. Parmi les principaux apports, je voudrais tout d'abord citer la pleine application du règlement dit Omnibus, ce que la France avait jusque-là refusé de faire en sous-transposant le droit européen. Ainsi, tous les contrats d'assurance couvrant au moins 20 % des pertes seront éligibles à une indemnisation de 70 % de la part de l'État. Je pense ensuite à l'inscription d'un budget annuel de 600 millions d'euros. souligner l'engagement de maintenir, dans la durée, le taux de franchise, le taux de subvention des contrats d'assurance et le seuil d'intervention de l'État par filière. Tout cela devait initialement être défini par voie réglementaire, privant l'ensemble des acteurs de visibilité sur la portée de la réforme. à l'incitation à la prévention et à la révision des principaux points bloquant le recours à l'assurance, notamment avec le choix de la moyenne la plus avantageuse pour le calcul des indemnités et la révision des critères de surfaces à couvrir. relève le pilotage du nouveau dispositif par la commission tripartite, associant État, agriculteurs et assureurs, laquelle consultera toutes les filières agricoles avant la remise de ses recommandations.

pour nos agriculteurs et nos agricultrices, avec des conséquences économiques trop souvent dramatiques. La gestion de ces risques relève d'une question de souveraineté alimentaire pour notre pays. Le sur le sujet étant problématique, une réforme était bienvenue. Cependant, comme nous l'avons déjà souligné en première lecture, nous nous inscrivons contre la logique même de ce texte, qui privilégie le recours à l'assurance privée pour faire face à ces risques climatiques. Ce choix d'un désengagement de l'État au profit du secteur assurantiel nous semble à la fois inéquitable et inefficace. Inefficace, parce que des décisions stratégiques pour notre agriculture, notre alimentation et nos territoires seront confiées à des acteurs privés, avec un encadrement qui nous paraît insuffisant. En témoignent les récentes annonces sur les augmentations de tarifs des contrats MRC. Inefficace, car très peu d'éléments viennent articuler véritablement l'assurance climatique avec le développement de pratiques agricoles sources de résilience comme la diversification des cultures, l'agroforesterie, les pratiques de préservation de la vie des sols, alors qu'il s'agit de nos premières garanties de prévention des risques. Cette trop faible incitation à la transition agroécologique se retrouve malheureusement dans bien d'autres politiques publiques, comme le plan stratégique national de la PAC, le plan France 2030 ou les choix budgétaires de soutien à la haute valeur environnementale (HVE) au détriment de l'agriculture biologique. La présente réforme est fondée sur un système rejeté par l'ensemble des acteurs de l'agroécologie, comme en témoigne la prise de position du collectif Pour une autre PAC contre le financement européen de l'assurance récolte. Cela n'est pas sans rappeler les politiques de gestion des risques sanitaires liés à la grippe aviaire qui se font, là aussi, contre les acteurs des systèmes agricoles durables, lesquels incarnent pourtant, nous en sommes convaincus, l'avenir de notre agriculture. En plus d'être inefficace, ce système est inéquitable : les objectifs de couverture assurantielle sont de 30 % seulement en 2030 pour les prairies et l'arboriculture, malgré un grand renfort de financements publics. Rappelons aussi qu'il n'existe tout simplement pas d'offre disponible pour de nombreux secteurs. Ce seront les exploitations les moins en difficulté, celles qui dégagent le plus de trésorerie, qui seront les plus aidées, tandis que les autres ne pourront bénéficier que d'une indemnisation au rabais. Certes, cette minoration nous est imposée par le droit européen, mais le Gouvernement ou la majorité sénatoriale n'hésitent pas à travailler au changement de la réglementation européenne lorsqu'elle ne les satisfait pas. Ce ne fut pas tout à fait le cas ici

Des avancées ont certes été concédées pour tenter de limiter le caractère inégalitaire du texte. Le rapporteur, dont nous saluons le travail, a obtenu un engagement sur un déclenchement de la solidarité nationale à 30 % de pertes pour les productions bénéficiant de peu d'offres assurantielles. Nous reconnaissons cette avancée. Nous nous réjouissons aussi des engagements formulés pour une réforme de la moyenne olympique. Pour autant, ce texte ouvre clairement la voie à une baisse de la solidarité nationale, dommageable à la fois pour les producteurs et pour le maintien de productions diversifiées sur le territoire. La proposition d'un fonds mutuel solidaire faite par plusieurs groupes de gauche et par des acteurs syndicaux agricoles n'a pu être véritablement discutée, ce que nous regrettons. Elle permettrait pourtant de créer un système plus équitable, piloté par l'État et les agriculteurs, tout en s'articulant un système de financement permettant de mettre à contribution les secteurs de l'amont et de l'aval agricole, qui restent aujourd'hui les plus profitables. Les difficultés actuelles lors des négociations des prix viennent encore une fois nous le rappeler : les agriculteurs restent les grands perdants de la chaîne de valeur. Enfin, ce texte présente un recul majeur, à savoir la modulation de la DJA en fonction de la souscription à un contrat d'assurance ou d'un diagnostic établissant une maîtrise des risques. Il aurait pu être pertinent d'inclure des modules sur la gestion des risques dans le parcours à l'installation, la mesure proposée complexifie les démarches, ce qui nous semble une grave erreur à l'heure du défi du renouvellement des générations. Pour toutes ces raisons,

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, si la question d'une protection des agriculteurs contre les risques climatiques est cruciale, nous pensons que ce projet de loi ne répond pas à cette urgence. Il n'y répond pas, car il s'enferre dans le choix de l'assurance privée, alors que nous savons que ce système assurantiel, promu depuis des années, ne fonctionne pas. Ainsi, malgré les niveaux croissants de subvention publique de l'État et de l'Union européenne à ces contrats d'assurance ces quinze dernières années, le recours à l'assurance récolte reste minoritaire. il est important de rappeler que toute nouvelle croissance des soutiens publics à l'assurance privée, qu'elle soit portée par l'État ou par un prélèvement complémentaire sur le second pilier de la PAC, risque de se faire au détriment non seulement des autres objectifs de soutien- je pense aux aides bénéficiant à la fois aux territoires et exploitations les plus fragiles, en zones défavorisées et de montagne -, mais aussi au détriment des mesures favorables à la transition agroécologique des modèles agricoles. Ainsi, encore une fois, aucune nouvelle perspective n'est offerte à un secteur économique secoué par la crise, dont la capacité à continuer à produire, à assurer la sécurité alimentaire et à prendre soin des espaces ruraux est pourtant vitale.

mais aussi pénaliser ceux qui n'auront pas souscrit d'assurance, puisqu'ils seront moins indemnisés par l'État et seulement en cas de pertes exceptionnelles.

qu'il bénéficiera à toutes et à tous, car les assureurs vont se mettre autour d'une table et feront preuve d'un comportement vertueux. On aimerait vous croire, mais l'histoire récente vous contredit,

Et Groupama confirme cette tendance, puisqu'elle souligne d'ores et déjà, compte tenu de l'évolution du changement climatique, que la baisse des primes n'est sans doute pas à l'ordre du jour. De plus, les garanties des productions non assurables, évoquées à l'article 3, feront l'objet d'un traitement à part dans la détermination des seuils d'intervention de l'État.

nous réitérons notre opposition à la gouvernance que vous proposez pour l'ensemble du secteur, qui tend à accorder beaucoup trop de place aux assureurs, au détriment de la représentation du monde agricole la Codar. Il est essentiel de définir un nouveau régime ambitieux capable de répondre aux enjeux et défis de demain : un régime public, solidaire et mutualisé, couvrant de façon universelle toutes les agricultrices et tous les agriculteurs. Au contraire, vous faites le choix de soutenir l'assurance privée et de réduire la part de l'intervention publique directe, raison pour laquelle nous voterons contre les conclusions de cette commission mixte paritaire. La parole est à M. Pierre Louault, pour le groupe Union Centriste.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, à regarder de près le code rural, on attend beaucoup de l'agriculture et de la politique publique qui la soutient assurer à la population l'accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, reconquérir la souveraineté alimentaire de la France ou encore concourir à la transition énergétique. J'y ajouterai l'enjeu de vitalité des territoires auquel contribuent aussi les exploitants agricoles. Tout cela impose de les aider à protéger leur production des aléas climatiques, mais pas seulement. En effet, on ne peut pas demander aux agriculteurs de remplir des missions d'intérêt général sans, en retour, leur garantir la solidarité nationale pour des risques qui les dépassent ... Tout cela n'exclut pas de les responsabiliser à la mise en oeuvre d'outils de prévention quand c'est possible, bien entendu. Aussi, je me réjouis de voir émerger une réforme des dispositifs de gestion des risques climatiques en agriculture. C'est un sujet que mon groupe suit de longue date. Je rappelle que le Sénat avait approuvé, en 2020, la proposition de résolution du groupe du RDSE visant à encourager le développement de l'assurance récolte. Nous sommes face à une urgence. Alors que plus personne ne conteste la récurrence et la violence des intempéries, on constate un taux de couverture assurantielle des exploitations globalement très insuffisant. Disons-le clairement, le coût des primes d'assurance est un frein. Un effort est donc attendu en direction du soutien aux primes. Le projet de loi vise à apporter une réponse à cet égard. Je citerai, notamment, la prise en compte du taux maximal proposé par le règlement Omnibus afin de subventionner davantage les primes.

le cumul des indemnités issues des contrats d'assurance et des indemnisations versées par les pouvoirs publics répond aussi à une attente forte. Avec le système actuel, il est difficilement acceptable de constater que les agriculteurs non couverts sont mieux indemnisés que des exploitants ayant assuré leur récolte Ces deux avancées sont importantes. Je tenais cependant à exprimer quelques regrets. Tout d'abord, je souhaitais rappeler qu'une majorité du RDSE est favorable à l'assurance récolte obligatoire, comme mon collègue Henri Cabanel l'a souligné en première lecture. Faute d'une mutualisation générale des moyens, et donc d'une couverture obligatoire du risque climatique, de nombreux agriculteurs ne pourront toujours pas s'assurer à un coût raisonnable. Ils seront ainsi en grande difficulté en cas de lourdes pertes de récolte. un mot, également, sur la question de la moyenne olympique, même si le texte a prévu une obligation de réflexion sur l'évolution de son mode de calcul. Comme vous le savez, monsieur le ministre, le système dit de la « moyenne olympique pour indemniser les pertes de récolte a été fixé par l'Union européenne sur la base des règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), mais tout cela date de 1994. Or, depuis, l'accélération du réchauffement climatique rend de plus en plus fréquentes les intempéries et les sécheresses, lesquelles affaiblissent les rendements agricoles et, par ricochet, minorent l'indemnisation des pertes. Enfin, nous souhaiterions vivement que soit réalisé, d'ici à trois ans, un bilan sur le taux de pénétration de l'assurance récolte afin de pouvoir corriger les faiblesses du nouveau système. Mes chers collègues, pour finir, la commission mixte paritaire a conservé un équilibre satisfaisant. Le RDSE approuvera ses conclusions, car ses membres sont attachés à la protection du travail, des investissements et surtout des

cours des cinq dernières années, les agriculteurs gardois, dans leur immense majorité, ont connu au moins trois sinistres. Malheureusement, je sais que beaucoup de mes collègues tirent exactement le même bilan dans leurs départements respectifs. Ce constat partagé en appelle un autre : face au changement climatique, notre gestion des risques en agriculture n'est plus à la hauteur ! Notre fonctionnement actuel fondé sur une articulation peu lisible entre le régime des calamités agricoles- dont sont exclues certaines cultures -et l'assurance privée ne permet pas, ne permet plus de sécuriser les agriculteurs français. Aujourd'hui, seulement 18 % de la surface agricole nationale est couverte par une assurance multirisque climatique. Ce simple chiffre illustre l'ampleur du problème auquel nous sommes confrontés.

et que notre excédent commercial agricole a tendance à diminuer depuis une quinzaine d'années, la question qui nous est posée est bien celle de notre souveraineté alimentaire. Monsieur le ministre, une réforme du système de l'assurance agricole était nécessaire et même urgente. Celle-ci est demandée, avec constance, depuis plusieurs années, par les sénateurs socialistes. Comme nous l'avons exprimé en première lecture,

L'application maximale du règlement Omnibus avec une franchise abaissée à 20 % et une subvention rehaussée à 70 % est un préalable important pour renforcer l'attractivité des contrats d'assurance. Monsieur le ministre, lors de nos derniers échanges, en réponse à un amendement de notre groupe, vous vous êtes engagés ici même à avancer sur la moyenne olympique. Il s'agit d'adapter ce référentiel, qui ne correspond plus à la réalité à laquelle sont confrontés nos agriculteurs.

doit nous conduire vers un système universel. C'est le coeur de la réforme et c'est un point fondamental pour les sénateurs. Malheureusement, le législateur n'a pas de visibilité sur l'offre assurantielle qui sera proposée aux agriculteurs. À nos yeux, il est indispensable que celle-ci soit véritablement attractive pour chaque filière. Aucun agriculteur ne doit être laissé de côté. Monsieur le ministre, avec ce projet de loi, vous avez choisi de confier cette responsabilité au prochain exécutif nous pouvons le regretter ... L'universalité de ce nouveau système dépendra néanmoins de la part de solidarité nationale qui accompagnera le dispositif. C'est dans ce cadre que le travail mené par le Sénat aura permis de renforcer considérablement le texte. Je remercie d'ailleurs notre collègue Laurent Duplomb de nous y avoir pleinement associés. En inscrivant un budget annuel de 600 millions d'euros et en définissant les seuils d'intervention de l'État à 50 % pour les cultures dites « assurables » et à 30 % pour les autres, nous avons donné du corps à ce qui est désormais un projet de loi d'orientation. Monsieur le ministre, votre projet de loi sort renforcé du travail parlementaire. Les chiffres sont souvent le nerf de la guerre. Or les chiffres qui ont été inscrits dans le texte issu de la commission mixte paritaire sont de nature à sécuriser les agriculteurs français à l'égard d'une réforme qui dépendra en grande partie de la confiance qu'elle sera en mesure d'inspirer au monde agricole. Cette confiance doit s'installer dans la durée et se travailler dès à présent. À ce titre, je me permets d'ouvrir une parenthèse pour rappeler qu'il est urgent de répondre efficacement aux attentes suscitées par le plan Gel de 2021. À ce jour, les agriculteurs que j'ai rencontrés sont encore dans le flou. Enfin, pour en revenir au texte, les améliorations qui ont été apportées permettront de renforcer le poids de l'engagement budgétaire de l'État en faveur de la résilience de notre agriculture, en prévision des prochains projets de loi de finances. en quelque sorte, monsieur le ministre, d'un service que nous vous avons rendu à vous et à votre ministère. Il est aujourd'hui indispensable de faire entendre, y compris au ministère des finances, que nos agriculteurs ont besoin de la solidarité nationale.

ma dernière intervention de la quinzième législature portera sur ce texte, qui vient clore le beau chapitre agricole de ce quinquennat. Et quel texte, mes chers collègues ! Le Premier ministre l'a souligné hier lors des questions d'actualité au Gouvernement, y voyant un changement complet de l'assurance récolte attendu attendu « depuis des années ». Selon un vieil adage, à quelque chose malheur est bon : en effet, le gel historique dramatique de l'année 2021 a contribué à la convergence de tous les acteurs. Le Président de la République et le Gouvernement ont alors pris la décision de mettre les bouchées doubles pour aboutir à une réforme systémique de notre modèle assurantiel. J'en profite pour saluer également votre action, monsieur le ministre, car vous avez été sur ce dossier un chef d'orchestre volontariste. Vous avez su imprimer un tempo accéléré pour que nos agriculteurs puissent prendre possession de cette réforme dès l'année prochaine. Je pense qu'ils vous en seront reconnaissants. un projet de loi dont les rouages doivent aussi beaucoup au député Frédéric Descrozaille. Il a été un rapporteur travailleur et passionné, puisqu'il n'a pas compté ses heures pour concilier des positions contraires. Il a su trouver à force d'écoute, mais aussi de détermination, le chemin des compromis salvateurs. Nous saluons ici son travail remarquable. Nous devons aussi apprécier l'intelligence collective de nos deux assemblées, qui ont su travailler sans arrière-pensée lorsque l'intérêt d'une cause commune était en jeu. Je remercie notre rapporteur, Laurent Duplomb, de son esprit de conciliation et je salue la complémentarité de ses travaux. travaux. Il aurait été tentant, à quelques semaines d'une échéance électorale majeure, de renverser la table par opportunisme politique, mais cela n'a pas été le cas. Chacun a su avancer sans esprit partisan. C'est pour moi un bel exemple d'unité réfléchie entre des adversaires politiques qui se respectent., tout le monde peut être satisfait des conclusions de cette même si, avec le recul, le résultat n'était pas gagné d'avance. Il est vrai que l'article 17 a surpris un peu tout le monde. Il est louable de rassurer nos agriculteurs par des éléments chiffrés leur donnant de la visibilité. C'est l'esprit de cet article. La convergence nous a donc amenés à écrire noir sur blanc et à inscrire dans le marbre les fondements chiffrés de cette architecture à trois étages. Je fais référence, par exemple, à la mention du budget annuel de 600 millions d'euros. Le texte qui nous est proposé reconnaît aussi l'importance de la concertation avec l'ensemble des parties prenantes, réunies au sein de la Codar. La commission devra ainsi discuter de la maîtrise budgétaire d'une telle réforme. L'ossature du monument qui est devant nous vient d'être finalisée, mais il reste encore beaucoup de travail. La consultation sera essentielle pour le projet de pool d'assureurs, une ambition nécessaire pour une plus grande transparence dans la constitution des prix, afin de proposer des assurances accessibles au plus grand nombre d'agriculteurs. Faisons confiance aux corps intermédiaires, aux organisations interprofessionnelles, aux assureurs pour continuer à porter cette réforme vitale qui vise à redonner confiance à nos agriculteurs. Quant à nous, nous nous retrouverons dès l'automne prochain, lors de l'examen de la prochaine loi de finances pour concrétiser dans le dur les engagements financiers de ce gouvernement. Mes chers collègues, soyons fiers de ce texte fondateur et ne boudons pas notre plaisir. Soyons fiers de ce quinquennat qui a su réparer notre agriculture. Notre groupe votera des deux mains ce texte historique très attendu. Nos agriculteurs comptent désormais sur nous pour les accompagner dans la révolution agroécologique. En attendant, je vous donne rendez-vous au Salon de l'agriculture ! Conformément

et permettant d'accéder à internet

le 17 février dernier, la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale ainsi que la commission des affaires économiques du Sénat sont parvenues à un accord unanime sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet. Je tiens à remercier vivement M. Bruno Studer de son esprit d'écoute et d'ouverture. Nous avons eu des échanges constructifs et complémentaires, qui nous ont permis d'élaborer un texte commun. Nous souhaitons toutes et tous une meilleure protection de la présence en ligne de nos enfants et de nos adolescents, dont la vie est de plus en plus virtuelle : c'est cet objectif qui nous a rassemblés. En tant que rapporteure, je m'étais fixé une feuille de route : je peux me féliciter aujourd'hui de sa tenue, car les apports et les principes posés par le Sénat ont tous été conservés. Nombreux sont les députés qui, mardi dernier, ont salué nos travaux ! Le texte que je vous propose d'adopter aujourd'hui demeure mesuré : il permettra de mieux accompagner les familles, d'encourager l'utilisation du contrôle parental, sans s'immiscer de façon excessive dans la relation intime qui lie les enfants à leurs parents. Ce texte est aussi adapté aux pratiques numériques de nos enfants et de nos adolescents, en ciblant les principaux appareils connectés utilisés aujourd'hui, qu'ils soient neufs ou reconditionnés, notamment les smartphones, les tablettes, les ordinateurs et les consoles de jeux. Le périmètre défini par l'Assemblée nationale était pertinent. Ce texte permet surtout de nouvelles avancées pour une meilleure protection de nos enfants et de nos adolescents sur internet. En commission, nous avions élargi le périmètre des contenus susceptibles de faire l'objet d'un contrôle parental, en retenant la notion « d'épanouissement » des personnes mineures. Un contrôle parental élargi, c'est davantage d'enfants et d'adolescents protégés. Tel est notre objectif principal. Nous avions également renforcé la protection des données à caractère personnel des mineurs. C'était un oubli du texte qui nous avait été transmis. Le sujet est pourtant central quand nous constatons que nos enfants et nos adolescents naviguent de plus en plus jeunes et de façon de plus en plus autonome sur internet, sans toujours être conscients de ce qu'ils acceptent ou de ce Je me félicite que ces deux dispositions importantes pour la protection de l'enfance et de l'adolescence demeurent inchangées. Ce texte a également été élaboré pour s'appliquer à l'état actuel du marché tout en prenant en compte les évolutions économiques et réglementaires qui doivent être anticipées à l'échelle de l'Union européenne. Sur ce point, la responsabilisation des fournisseurs de systèmes d'exploitation était une priorité de notre commission. Quand nous parlons de contrôle parental, il ne faut pas oublier qu'il s'agit avant tout d'une fonctionnalité logicielle et non d'un composant électronique assemblé par le fabricant. Nous avons travaillé à une rédaction commune permettant de prendre en compte la diversité des modèles économiques, notamment le fait que les fabricants sont aussi fournisseurs de systèmes d'exploitation. Nous avons souhaité que les responsabilités de chaque acteur soient bien identifiées, sans privilégier un modèle économique plutôt qu'un autre c'était indispensable pour que cette proposition de loi soit pleinement opérationnelle. En ce qui concerne la commercialisation du matériel sans système d'exploitation, le Sénat a explicitement abordé en séance publique une question qui avait été écartée.

Sur la question de la désinstallation, là encore, le Sénat a introduit dans le débat un sujet qui avait été mis de côté. La désinstallation doit être gratuite pour l'utilisateur lorsqu'elle est techniquement possible, ce qui n'est pas toujours le cas. Nous avons trouvé un équilibre entre les contraintes des acteurs économiques et la nécessité de faire progresser les droits des utilisateurs ; il s'agissait d'une préoccupation également importante pour notre commission.

Cet article vise à conditionner l'entrée en vigueur du texte à la réponse de la Commission européenne attestant de sa conformité avec le droit de l'Union. Il y a deux jours, le texte a de nouveau été notifié à la Commission européenne, conformément à notre souhait initial et à l'engagement de M. Studer, que je remercie encore.

Madame la présidente, madame la présidente de la commission des affaires économiques, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, je remercie tout d'abord l'ensemble des sénateurs et députés qui ont permis d'aboutir à ce texte de qualité et d'équilibre. Je veux reprendre, ici, les mots d'Adrien Taquet à la tribune de l'Assemblée nationale mardi soir : il rappelait que la protection de l'enfance est un continuum dont les activités en ligne ne forment qu'une partie.

Évidemment, les parents jouent un rôle central dans ces apprentissages. Grâce à vos travaux, nous pouvons estimer que ceux-ci seront mieux équipés pour accompagner leurs enfants dans leur vie en ligne. Ils devront donc choisir d'activer ou non le contrôle parental lorsqu'ils installent un nouveau terminal pour leurs enfants. Je suis convaincu que rendre explicite ce choix permettra d'augmenter significativement l'usage de ces systèmes de contrôle parental sur les terminaux utilisés par les mineurs. Lors de l'appel lancé le 11 novembre dernier, dans le cadre du Forum de Paris pour la Paix, en faveur de la protection de l'enfance en ligne, le Président de la République avait notamment mis l'accent sur l'importance d'un meilleur usage des systèmes de contrôle parental. Cette nouvelle obligation s'inscrit en cohérence totale avec cet appel. De façon plus générale, le Gouvernement est engagé depuis plusieurs années pour la protection de l'enfance en ligne. Nous en avons fait une de nos priorités d'action. Cette proposition de loi s'insère donc dans une politique plus large de protection de l'enfance des pouvoirs publics dans l'environnement numérique. Je pense à la lutte conte le cyberharcèlement, qui touche notamment les enfants et les adolescents à une période charnière où ils peuvent être particulièrement vulnérables. Je pense au protocole d'engagement afin de limiter l'exposition des mineurs à la pornographie en ligne, qui a notamment mené à la création du site « jeprotegemonenfant.gouv.fr

Je pense à la prise en compte des spécificités des utilisateurs mineurs dans les projets de régulation des plateformes au niveau européen. Il s'agit, notamment, du, dont la France mène actuellement les négociations en trilogue

le Gouvernement s'est engagé et s'engage avec constance et détermination pour protéger les enfants et les adolescents dans leur vie numérique. Je rappelle, à ce titre, deux chiffres terribles : près d'un parent sur trois n'a pas connaissance des outils de contrôle parental, alors que trois parents sur quatre adhèrent à l'idée de l'usage d'un tel outil Les parents sont donc demandeurs de ces outils. Cette proposition de loi permettra à chaque parent de saisir facilement l'occasion de les activer. Sur le plan technique, les amendements et améliorations successives votés au cours des différentes lectures de ce texte ont permis d'apporter des éclaircissements utiles et salutaires. Vous avez précisé le rôle des différents acteurs de la chaîne de valeur et de commercialisation, détaillé le contenu du décret prévu par l'article 1, affiné le champ d'application et explicité certains cas particuliers, notamment la gestion des terminaux reconditionnés et de ceux qui sont vendus sans système d'exploitation. Ces ajouts et ajustements apportent des clarifications utiles et permettent d'aboutir à un texte à la fois équilibré et ambitieux. Cette proposition de loi permettra d'empêcher les enfants d'accéder à des contenus préjudiciables et assurera un socle minimal de fonctionnalités accessibles sans surcoût. Elles seront présentes sur tous les terminaux pour protéger les utilisateurs mineurs. Je rappelle, par ailleurs, que l'esprit de cette proposition de loi porte plus loin : elle permettra, je l'espère, aux parents d'engager une discussion positive avec leurs enfants sur les pratiques numériques, ainsi que sur les opportunités et les dangers de leurs usages. Telle était très largement la volonté de Bruno Studer, président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, lorsqu'il a

La puissance publique doit créer les conditions de la confiance, de l'« encapacitation » et de l'information des parents pour que ceux-ci puissent jouer leur rôle d'éducateurs éclairés. Nous devons leur proposer des outils pertinents et bienvenus au moment clé qu'est l'accès de l'enfant à son premier smartphone ou à sa première tablette. Ainsi, en donnant aux parents un outil supplémentaire pour accompagner leurs enfants, cette proposition de loi s'inscrit en complète cohérence avec l'action de ce gouvernement. cette discussion a pu être menée et salue particulièrement le travail de Mme la rapporteure. J'espère que nous pourrons renouveler et poursuivre ce combat pour la protection de l'enfance en ligne.

le sujet de la protection des mineurs sur internet est un véritable enjeu de société. Nos enfants grandissent dans un environnement numérique, sont des utilisateurs naturels et deviennent de plus en plus jeunes des consommateurs intensifs des nouvelles technologies. et des libertés (CNIL), datant de 2020, dresse un constat édifiant et témoigne également de deux grandes tendances : le souhait des mineurs de gagner en autonomie sur internet des parents de renforcer leur protection en ligne. Cette étude fait apparaître que la navigation sur internet sans intervention parentale est généralisée : 82 % des enfants de 10 ans à 14 ans vont régulièrement sur internet sans leurs parents

Ils sont ainsi exposés très tôt à une multiplicité de risques : cyberharcèlement, mauvaises rencontres, exploitation des données personnelles, exposition à des contenus haineux, violents, pornographiques. Sur ce dernier point, des études montrent que près d'un tiers des enfants de 12 ans ont déjà été exposés à des contenus de ce type, souvent de manière involontaire en naviguant sur le Net.

Qui plus est, quand ils installent cet outil, ils ne le font souvent que sur un seul appareil. Or les jeunes utilisent en moyenne quatre écrans différents par jour. C'est dire combien il est nécessaire de mieux protéger nos enfants et nos adolescents sur internet, et de faciliter l'utilisation du dispositif de contrôle parental. Comme l'a souligné Mme la rapporteure, Sylviane Noël, dont je veux saluer le travail, ce texte est opportun, mais son ambition était initialement limitée. Si l'installation du contrôle parental sur les équipements semble généralisée, cette situation ne repose que sur la volonté des leaders sur un marché très concentré. Inscrire dans la loi l'obligation d'équiper les outils donnant accès à internet d'un système de contrôle parental aisément accessible et compréhensible, dont l'activation devra être proposée lors de la mise en service de l'appareil, permettra de sécuriser la protection des mineurs.

il a renforcé la protection des données personnelles des mineurs collectées lors de l'activation du dispositif de contrôle parental. C'était un aspect complètement absent de la proposition de loi

Cinquièmement, nous avons voulu éviter les effets de bord, notamment pour les ordinateurs commercialisés sans systèmes d'exploitation à des fins professionnelles ou à des particuliers.

C'est pourquoi le groupe Les Républicains votera pour le texte issu de l'accord trouvé en commission mixte paritaire. La parole est à M. Thomas Dossus, pour le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui en deuxième lecture traite de la protection des enfants face à des contenus violents, pornographiques et haineux sur internet, ce qui est loin d'être anecdotique. Le texte se trouve à l'intersection de plusieurs sujets d'importance comme le libre accès à internet, la nécessaire protection des enfants, la liberté des choix éducatifs ou encore la protection des données. Son objectif principal est simple prévoir la présence d'un dispositif de contrôle parental préinstallé sur les terminaux permettant l'accès à internet. Le fonctionnement du dispositif, ses spécificités techniques, le nécessaire contrôle de l'application de la mesure, la certification, tout cela est renvoyé à un décret en Conseil d'État. Je me réjouis que la navette ait utilement enrichi ce texte. Elle a permis d'ajouter en première lecture la nécessaire protection des utilisateurs des terminaux pour que leurs données ne soient ni commercialisées ni utilisées à des fins de marketing, ce qui est loin d'être un détail, car nous connaissons l'avidité des Gafam pour ces précieuses données et leur ingéniosité à utiliser tous les moyens possibles pour les collecter. Je me réjouis également que nos amendements concernant les terminaux vendus sans système d'exploitation, qui avaient été rejetés au Sénat, aient finalement été repris en commission mixte paritaire.

Nous saluons également le fait que le texte consacre la liberté des utilisateurs de désinstaller le logiciel de contrôle parental s'ils n'en ont pas l'usage. Là encore, la mesure n'a rien d'anecdotique, puisque maintenir une couche logicielle inutile sur un smartphone consomme de la mémoire, réduit l'usage qui peut en être fait et,, influence grandement la décision de l'utilisateur L'impact environnemental des pratiques numériques provient majoritairement de la consommation indécente des matières premières, en particulier des terres rares, nécessaires pour fabriquer nos appareils. Tout ce qui permet de prolonger la durée de vie des terminaux est donc une avancée. Vous l'aurez compris, nous voterons pour cette proposition de loi,

Non, la promesse naïve du progrès numérique sans limites, de l'innovation forcément vertueuse des licornes ne doit pas être le fondement de notre politique éducative. Il est nécessaire de développer l'esprit critique de la jeunesse à l'égard du numérique. En effet, comment utiliser internet, quel contenu éviter, quelle exposition aux écrans autoriser ? Comprendre et déconstruire le fonctionnement des algorithmes, lutter contre la désinformation et le harcèlement, tout cela s'apprend. Faire entrer non seulement le numérique à l'école, mais aussi le questionnement sur ses usages, ses dangers et ses limites, voilà qui devrait être un objectif partagé par tous. Ce que nous voulons, c'est l'éducation populaire au numérique. La parole

et qui illustre la place croissante que prennent internet et les outils numériques dans notre quotidien, de manière toujours plus précoce. Si le contrôle parental n'est pas une solution miracle, il est néanmoins un outil utile pour réduire le risque d'accéder à des contenus inappropriés, voire dangereux, ce qui se produit souvent de manière involontaire pour les plus jeunes. Aujourd'hui, un nombre trop important de parents sont démunis % des enfants de 6 à 10 ans sont protégés par un outil de contrôle parental, et encore, pas sur l'ensemble des équipements qu'ils utilisent. Cette proposition de loi qui vise à faciliter l'usage du contrôle parental est donc bienvenue.

le risque d'altérer la relation de confiance entre les parents et le mineur [ ...] ; le risque d'entraver le processus d'autonomisation du mineur [ ...] ; le risque d'habituer le mineur à être sous surveillance constante. » Toutefois, comme Toutefois, comme nous l'avions dit en première lecture, les enfants ne sont pas des utilisateurs comme les autres. À ce titre, plus ils sont jeunes, plus ils doivent être protégés et informés face à la multiplication de contenus dangereux ou inappropriés. Pornographie, violence, contenus haineux, cybermalveillance, jeux d'argent, la liste des contenus pouvant avoir un effet délétère sur les enfants et les adolescents est toujours plus importante. Le modèle économique d'internet étant basé sur la rétention de l'attention, la publicité, donc l'audience, conduit à ce que ces contenus soient de plus en plus faciles d'accès et gratuits. De la même manière, les mineurs doivent être protégés d'une exposition trop importante aux écrans, elle-même addictive. Il s'agit non seulement d'une question sociétale majeure, mais aussi d'un enjeu de santé publique. De plus, le Sénat a insisté sur la nécessité de protéger les données personnelles des mineurs. Ce sujet est central tant les enfants font l'objet d'un ciblage publicitaire et de techniques de marketing féroces. Certes, la loi ne réglera pas tout ; il est indispensable d'encourager les actions de prévention, notamment en milieu scolaire, et de mettre en oeuvre une démarche globale d'accompagnement des usages numériques des enfants, en particulier autour des contenus. Toutefois, nous pensons que les travaux de nos assemblées ont produit un texte équilibré, permettant un meilleur accompagnement des familles. C'est pourquoi nous voterons en faveur des conclusions de cette CMP et nous saluons le travail de Mme la rapporteure. La parole

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, lors de la séance du 9 février 2022, le Sénat a voté les apports de notre commission des affaires économiques sur la proposition de loi visant à encourager l'usage du contrôle parental sur internet. L'équilibre trouvé et validé dans le cadre de la commission mixte paritaire reprend les principales avancées du Sénat : nous pouvons nous en féliciter. J'ai l'honneur de faire partie de cette assemblée depuis seulement quelques semaines. Il s'agit de ma première expérience comme chef de file pour le groupe Union Centriste, et ce sur un texte dont le sujet est majeur, puisqu'il s'agit de la protection des enfants face aux dangers du numérique. L'enjeu dépasse l'esprit partisan et je me réjouis d'avoir assisté à un travail collaboratif et constructif avec les députés et le Gouvernement. Je remercie en particulier notre rapporteure Sylviane Noël d'avoir porté nos réflexions communes. Les apports du Sénat ont été substantiels. De manière synthétique, j'en citerai quelques-uns, notamment l'interdiction d'utiliser les données personnelles des enfants à des fins commerciales, ce qui est essentiel pour leur protection l'intégration de l'amendement de notre collègue Catherine Morin-Desailly visant à prévenir le danger à la surexposition précoce des enfants aux écrans ; la garantie de pouvoir acquérir sur le marché des équipements dits

Le contrôle parental sera donc un outil supplémentaire pour protéger nos enfants des dangers de l'internet. Je souhaite accompagner nos travaux d'une réflexion

que, « quand un écran s'allume, un enfant s'éteint ». Oui, plus de 5 000 études prouvent que la présence d'objets connectés a des effets délétères sur les tout-petits. Elles démontrent ainsi que le cerveau, lorsqu'il est privé des bonnes stimulations, peine à créer de bonnes connexions cérébrales. Les appareils à écran dans l'environnement de l'enfant, y compris ceux des parents

ou de motricité. Les pédopsychiatres et les infirmières scolaires tirent la sonnette d'alarme depuis des années, tant ils relèvent d'effets néfastes accrus sur les enfants soumis à la violence des images ou des vidéos.

Comme je le développais dans ma précédente intervention, au-delà des sites déjà existants de sensibilisation des parents, l'accompagnement pédagogique de l'enfant est essentiel. Il

celle de réévaluer et de repenser le dispositif du « permis internet », déjà expérimenté en classe de CM2, et de le rendre obligatoire afin de former nos enfants à l'éducation numérique dès le primaire. une fois votée, s'appliquera dans un cadre ciblé, il sera également nécessaire de sensibiliser et de développer le sens critique de nos enfants à l'égard de nouvelles technologies extrêmement évolutives, tels les robots et l'intelligence artificielle.

disposera-t-elle de tous les moyens nécessaires ? Enfin, la question de la protection des enfants et de la stratégie employée pour cela doit bien évidemment se poser au niveau européen. Du fait de la libre circulation des biens et des personnes, il paraît essentiel d'harmoniser ce type de mesures au niveau de l'Union européenne. un sujet de plus à traiter dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Le groupe Union Centriste se félicite toutefois du pas franchi aujourd'hui et votera ce texte. La parole

concilier la neutralité du web et la protection des mineurs face aux dangers de la toile, tel était l'objectif de cette proposition de loi et je me réjouis de l'issue conclusive de la commission mixte paritaire. Lors de la première lecture, j'avais insisté sur plusieurs éléments d'abord sur la forte présence des 11-14 ans sur internet et sur les multiples possibilités de contourner le contrôle parental- nous ne réglerons pas cela aujourd'hui

Cet état de fait, nous le constatons et nous le dénonçons depuis de nombreuses années sur ces travées, sans toutefois trouver de solution miracle pour y remédier et protéger nos adolescents. En ce qui concerne l'effectivité de cette proposition de loi, je le répète, le droit ne peut pas tout. La lutte contre les différentes dérives d'internet n'est possible qu'avec davantage de moyens accordés à la sensibilisation des parents comme des enfants.

Nous saluons la bonne tenue de cette CMP, qui a permis de conserver en grande partie la rédaction du Sénat, notamment sur l'amélioration des dispositifs de prévention des fabricants à destination des usagers ou sur la protection des données personnelles des mineurs. Au sujet de l'accessibilité du dispositif, rappelons que c'est la principale condition de sa réussite. La gratuité prévue à l'article 3 est donc bienvenue : toute personne qui souhaitera se saisir du dispositif pourra ainsi en bénéficier. Finalement, nous aboutissons à un texte équilibré, qui responsabilise aussi bien les fournisseurs des systèmes d'exploitation que les fabricants, tout en garantissant les droits des consommateurs. Il nous reste donc à attendre le verdict de la Commission européenne quant à sa conformité au droit de l'Union européenne et au principe du bon fonctionnement du marché intérieur. La période que nous connaissons et les élections à venir doivent nous mobiliser dans la lutte contre la propagation des contenus haineux et des, en particulier contre les effets qu'ils peuvent avoir sur les plus jeunes.

paritaire. La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

particulièrement pertinente au regard des évolutions technologiques des terminaux qui sont aujourd'hui à la disposition de nos enfants mineurs et de leurs usages. Je rappellerai ici deux chiffres : 92 % des 12-17 ans ont un téléphone portable,

ne doit pas se substituer à la discussion avec les adultes responsables sur les dangers d'un temps d'écran trop long et de la consultation de contenus dérangeants, voire malveillants, il reste nécessaire que des réglages et des logiciels y contribuent. La présente proposition de loi prévoit que les équipements ou services permettant d'accéder à internet fassent l'objet d'obligations renforcées afin de rendre plus systématique, simple et convivial l'usage par les parents des dispositifs de contrôle. Elle est adaptée aux pratiques numériques de nos enfants et de nos adolescents. Elle cible une grande diversité d'appareils qui permettent d'accéder à internet, qu'il s'agisse des smartphones, des tablettes, des ordinateurs, des consoles de jeux vidéo ou de certains objets connectés, tout en incluant les appareils reconditionnés. Nos échanges au Sénat ont permis de répondre à plusieurs interrogations. La question de la commercialisation des équipements sans système d'exploitation a été soulevée. Une précision utile, qui a permis de clarifier le sujet, a été apportée et cette commercialisation demeure possible.

La désinstallation doit être gratuite pour l'utilisateur lorsqu'elle est techniquement possible, ce qui n'est pas toujours le cas, notamment lorsque le contrôle parental est directement intégré dans les paramètres. Dans le cas où le fabricant est aussi le fournisseur du système d'exploitation, il lui appartient d'intégrer un dispositif de contrôle parental à ses équipements terminaux. En revanche, lorsqu'il sous-traite entièrement cette tâche à un tiers, alors il semble logique que ce tiers soit responsable de l'intégration d'un tel dispositif. Il certifiera alors au fabricant que son système d'exploitation est conforme à la loi, à charge pour ce dernier de communiquer ce certificat aux autres acteurs de la chaîne économique. Dans son habituelle sagesse, le Sénat a souhaité que les fabricants contribuent à la diffusion de l'information disponible sur les risques liés à l'exposition précoce des enfants aux écrans. mesure fait reposer une obligation somme toute modérée, mais très utile sur les fabricants, dès lors que celle-ci ne se traduit pas par un marquage de l'ensemble des appareils vendus en France, ce qui ne serait pas conforme au droit de l'Union européenne. outre, le Sénat a renforcé la protection des données à caractère personnel des personnes mineures. Le sujet est important, car nos enfants et nos adolescents naviguent de plus en plus jeunes et de façon de plus en plus autonome sur internet, sans toujours être conscients de ce qu'ils acceptent. Enfin, Enfin, l'article 3 , introduit par le Sénat, conditionne l'entrée en vigueur du texte à la réponse de la Commission européenne attestant sa conformité avec le droit de l'Union européenne. Le texte final sera donc de nouveau notifié à la Commission européenne afin de s'assurer de sa compatibilité avec le bon fonctionnement du marché intérieur. au nom de l'intérêt de l'enfant, de sa protection et de celle de l'adulte qu'il deviendra, les élus du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain se félicitent de l'issue donnée par le Parlement à cette proposition de loi. Ils voteront en faveur des conclusions de cette CMP.

La toile multiplie les contenus et interactions directement accessibles aux plus jeunes. Il ne s'agit pas ici de mettre fin à certains contenus haineux ; cela sera l'objet de défis à venir. À cet égard, les travaux de la députée Laetitia Avia doivent nous inspirer. de loi peut s'assimiler à une clé transmise aux parents pour interdire, s'ils le souhaitent, certains accès à leurs enfants. Sur ce point, elle apporte des réponses salutaires. Les modalités d'approche conviennent tant à nos collègues députés qu'au Sénat, dont les apports ont d'ailleurs été nombreux et bénéfiques. J'en profite pour saluer les travaux transpartisans de notre rapporteure, élaborés dans des temps particulièrement contraints. Comme vous le savez, ce texte impose que soit proposée l'activation d'un contrôle parental lors de la mise en service des terminaux permettant d'accéder à internet.

impossible d'évoquer la régulation du numérique sans évoquer le droit communautaire. Nous devons nous assurer que ce texte est bien compatible avec la législation européenne. Or une telle notification, effectuée après son dépôt à l'Assemblée nationale, pouvait paraître prématurée.

Pour conclure, notre groupe salue l'atterrissage en douceur de cette proposition de loi utile et gage de sécurité pour les parents. comme l'a très bien indiqué Bruno Studer, ce texte « ne remplacera jamais le rôle des parents dans le dialogue et la compréhension à l'égard de leurs enfants. »

tout en leur permettant de continuer à profiter des possibilités que leur offre cette technologie. Une autre proposition de loi que nous avons examinée aujourd'hui visait à renforcer la cybersécurité des Français en imposant la publication des résultats du diagnostic de sécurité. Nous avons amélioré l'information

En 2019, une étude démontrait qu'en moyenne les enfants détenaient un smartphone dès l'âge de 10 ans. Compte tenu du développement intensif des technologies numériques, celui-ci devient une porte d'accès facile au vaste espace que constitue internet.

Or nous savons bien que l'accès précoce et non préparé à la pornographie peut emporter des conséquences très graves sur la vie affective et sexuelle de nos adolescents.

celui-ci activé, les jeunes internautes ne pourront plus consulter des contenus susceptibles de leur porter préjudice. Cette fonctionnalité sera disponible sur tous les appareils, y compris ceux vendus d'occasion. Nous donnons ainsi des moyens aux parents de mieux protéger leurs enfants : à eux de s'en saisir. En effet, il reviendra aux parents d'activer la fonction de contrôle parental sur les dispositifs utilisés par leurs enfants. l'initiative du Sénat, le texte précise en outre que les données personnelles recueillies lors de l'activation de cette fonction ne pourront pas faire l'objet d'une exploitation commerciale. Ce texte constitue donc une étape supplémentaire visant à faire d'internet un espace civilisé et régulé. D'autres lois, notamment européennes, sont en cours de préparation. Ce travail est indispensable pour garantir la liberté et la sécurité de nos concitoyens dans le cyberespace. et Territoires est très attaché à ce qu'internet soit soumis aux mêmes règles que les autres espaces de notre République. Nous voterons donc en faveur de l'adoption de cette proposition de loi. Permettez-moi de conclure en saluant le travail de Mme la rapporteure.